Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, hier, l'épidémie de la covid-19 causait 292 décès supplémentaires, nous rapprochant encore davantage de la barre redoutée des 100 000 morts. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux soignants, épuisés. Un an après, le virus est toujours là, mais la résilience des citoyens, la force de nos professionnels de santé et l'engagement des élus s'efforcent de lui faire face. Le Premier ministre a ainsi annoncé des mesures spécifiques dans seize départements la semaine dernière. Elles sont nécessaires pour répondre aux appels des professionnels de santé submergés. Elles sont nécessaires, aussi, pour nous adapter à ce virus, qui mute et qui nous impose de modifier nos certitudes. les mesures de l'année passée ne sont plus celles d'aujourd'hui et ne seront probablement pas celles de demain. Elles peuvent dorénavant être territorialisées, comme à Mayotte, et variées, pour répondre aux besoins sanitaires sans oublier la santé mentale. Un an après, la covid rythme encore nos journées, mais une certitude est aujourd'hui acquise : la vaccination, sur tout le territoire, dans l'Hexagone comme en outre-mer, est notre unique issue. En un an, les scientifiques ont réalisé des prouesses, suspendant leurs recherches pour se concentrer sur un seul virus afin de développer des vaccins aux taux d'efficacité inégalés.

Pour autant, encore trop de personnes âgées ne parviennent pas à trouver de places pour se protéger, et la confiance à l'égard de certains vaccins continue d'être ébranlée par quelques cas isolés, mais inquiétants. Monsieur le secrétaire d'État, alors que la fatigue prend de plus en plus le pas sur la résilience, les citoyens ont besoin d'un horizon clair vers une sortie de crise. Quelles perspectives pouvez-vous nous apporter pour assurer la vaccination sécurisée de tous les Français qui le souhaitent, sur l'ensemble du territoire ?

à cette crise qui met notre système de santé à l'épreuve. Nous saluons de nouveau leur dévouement, ainsi que la résilience, que vous avez évoquée, de l'ensemble de nos compatriotes. Face à cette situation changeante, le Gouvernement adapte sa stratégie en concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment les élus locaux, avec pour seul objectif de rester le plus efficace dans cette lutte contre l'épidémie et de prendre les bonnes dispositions au bon moment. Vous avez justement noté que ces mesures sont de plus en plus territorialisées, car si le taux d'incidence et la pression hospitalière sont très élevés à certains endroits du territoire- je pense évidemment à l'Île-de-France et aux Hauts-de-France -, ce n'est heureusement pas le cas dans toutes nos régions. Nous avons choisi de prendre des mesures de freinage fortes dans seize départements à ce stade.

que nous souhaitons tous voir s'intensifier. Les vaccins sont le principal espoir de sortie de crise. Nous le répétons sans cesse : il faut vacciner et il faut se faire vacciner. Cela vaut pour l'outre-mer, évidemment, et cela vaut pour Mayotte, où 75 % des doses livrées ont été inoculées. Il faut néanmoins accélérer. La mobilisation de tous doit être totale, notamment celle des élus locaux. Je salue d'ailleurs votre engagement, monsieur le sénateur, à cet égard. Nos objectifs restent inchangés : vacciner 10 millions de Français à la mi-avril et 20 millions à la mi-mai. Le Président de la République, pour ce faire, a annoncé hier, vous l'avez entendu, que dès samedi prochain la vaccination sera élargie aux plus de 70 ans sans comorbidités. Pour n'oublier personne, l'assurance maladie appellera tous les plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinés afin de leur proposer un créneau. Des campagnes de vaccination ciblée seront enfin bientôt lancées,

Il y a un an, jour pour jour, la France entrait de nouveau dans l'état d'urgence. La soudaineté du premier confinement a pleinement justifié les difficultés d'organisation des élections municipales. un état d'urgence vise, par définition, à répondre aux urgences. Il ne doit pas affecter de façon déraisonnable des rendez-vous démocratiques planifiés de longue date.

ne nous y trompons pas : le conseil scientifique rendra un avis qui sera fonction des moyens et des innovations mis en oeuvre pour permettre le bon déroulement de ces élections. Ma question est simple, madame la ministre quelles propositions d'organisation de notre vie démocratique pouvez-vous mettre en avant pour faciliter une réponse positive du conseil scientifique à la tenue de ce temps fort de notre démocratie ?

Monsieur le sénateur Mickaël Vallet, je répondrai très clairement à la question que vous posez. Je le ferai d'autant plus volontiers que j'ai eu le plaisir et l'honneur de représenter le Gouvernement ici même pendant plusieurs heures, quand nous avons débattu,

Le Gouvernement, comme il s'y était engagé, a d'ailleurs immédiatement publié dès le mois de mars le décret de convocation des électeurs pour les 13 et 20 juin prochain. Dans cette loi que nous avons discutée et que vous avez votée, il est également fait mention du rapport du rapport du conseil scientifique, qui doit être présenté et transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 avril. À l'heure actuelle, nul ne dispose du contenu du rapport du conseil scientifique,

en lien avec les maires et les collectivités, à un protocole sanitaire strict, qui réponde à toutes les mesures que vous avez votées, notamment la mutualisation des fonctions d'assesseur et de président de bureau de vote.

M. Mickaël Vallet, pour la réplique. J'entends bien, madame la ministre, que les élections doivent se tenir « quoi qu'il en coûte », selon l'expression consacrée.

le vote par correspondance, l'étalement du vote sur trois jours, et j'en passe ! Le Gouvernement a rejeté toutes ces innovations démocratiques, qui valaient pourtant bien les grands débats de 2019 et la Convention citoyenne de 2020.

qui a rassemblé sous votre présidence plusieurs de vos ministres, le président du Sénat et les présidents des groupes de la Haute Assemblée, je vous ai demandé, au nom du RDSE, de retarder le début du couvre-feu de dix-huit heures à vingt heures, en raison de l'allongement de la durée du jour et de l'arrivée de l'heure d'été.

Pour les seize départements les plus touchés par la pandémie, vous avez ensuite annoncé une troisième variante de confinement, une troisième voie, à savoir un confinement « moins confiné », toujours vigilant dans l'espace privé, mais plus large dans l'espace public, permettant aux habitants de se déplacer davantage que lors des précédents confinements. Toutefois, c'était sans compter samedi sur la fameuse attestation dérogatoire de deux pages,

et la fatigue de nos concitoyens, mis à rude épreuve depuis un an. Monsieur le Premier ministre, en cas d'aggravation de la pandémie, quelles mesures envisagez-vous de prendre dans les seize départements de la zone rouge et dans ceux de la zone verte ? La parole est à M. le Premier ministre.

que j'organise de manière régulière avec les présidents des différents groupes du Sénat, comme du reste de l'Assemblée nationale, avant toute prise de décision. Je vous remercie également d'avoir observé que, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là,

que nous maintiendrons cette stratégie autant que cela sera possible. Il n'a échappé à personne, sur aucune travée de cette assemblée, que nous sommes face à une troisième vague particulièrement virulente.

durcir, en fonction de l'évolution de la pandémie, car nous avons le devoir de nous adapter, comme nous l'avons toujours fait ! Nous tenons également compte de ce que nous avons appris

conséquent, nous avons intégré cette considération dans les mesures prises, ce qui ne signifie pas, je le dis de façon très solennelle devant le Sénat, qu'à l'extérieur on puisse faire n'importe quoi

citer les propos des responsables de l'académie de Créteil : « Il y a eu un véritable tsunami de remontées de cas positifs par les écoles à traiter cette dernière semaine. Tous les médecins de l'éducation nationale du département sont sur le pont,

donc on mélange les élèves pour poursuivre l'accueil, au mépris du protocole sanitaire. Il n'y a pas de moyens de protection des personnels enseignants ou éducatifs pourtant en première ligne.

en cette période si particulière, nous avons deux responsabilités. La première est d'assurer la protection de nos élèves et de nos personnels. La seconde est de garantir la réussite scolaire. la protection de nos élèves et de nos personnels, je vous rappelle que nous avons déployé des protocoles sanitaires que nous ne cessons d'adapter. Vous avez évoqué, madame la sénatrice, la question des remplacements. Oui, il y a des remplaçants

200 000 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité dans nos établissements qui oscille entre 0,3 % et 0,5 %.

bovine. En 2020, alors même que les ventes de viandes bovines françaises ont progressé, le prix payé aux éleveurs n'a cessé de chuter, pour aboutir à un résultat particulièrement alarmant. Selon la Fédération nationale bovine, les éleveurs ont dû vivre avec moins de 700 euros par mois l'année dernière. La France est pourtant le premier producteur européen de viande bovine, avec 485 000 emplois qui contribuent à l'animation de nos territoires et façonnent nos paysages. La viande rouge représente 63 % de la viande consommée en France et fait partie intégrante de notre patrimoine gastronomique. Nous ne pouvons pas regarder sans réagir nos éleveurs disparaître en raison de prix inexplicablement bas, à l'image du cours des jeunes bovins. Nous ne pouvons pas laisser les éleveurs continuer de vendre leurs animaux à un prix inférieur d'environ un euro du kilogramme à leur coût de production, un coût de production qui ne cesse d'ailleurs La crise des éleveurs est accentuée par l'augmentation des prix des matières premières nécessaires à l'alimentation du bétail, ravivant ainsi des tensions sur le partage de la valeur ajoutée. loi Égalim, porteuse d'espoirs, censée rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs et grande distribution, tarde à porter ses fruits. agricole commune, la PAC, les inquiétudes se font grandes. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour soutenir concrètement et dans la durée l'élevage français, pour lui redonner de nouvelles perspectives ?

L'UNEF a donc désormais comme critère la couleur de peau dans ces réunions dites « racisées », mais pas « racistes » ! Hélas, ce syndicat n'en est pas à un coup d'essai. En 2019, il a tenté d'empêcher une représentation de la pièce d'Eschyle et a considéré l'émotion ressentie par les Français lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris comme « un délire de petit blanc ». On pourrait parler aussi de la récente affaire de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Aujourd'hui, l'arsenal juridique français permet de sanctionner toutes les formes de discriminations, particulièrement lorsqu'elles se fondent sur l'origine et la couleur de la peau. Le délit de provocation à la discrimination existe. Pourquoi n'y faites-vous pas référence ? Qu'attendez-vous pour simplement appeler à l'application de la loi pénale ? Au-delà de l'action judiciaire, chaque année, l'UNEF perçoit une subvention de 600 000 euros de l'État. Aussi, l'État doit-il continuer à financer l'organisation de réunions « racisées »

ces réunions se tenaient apparemment à l'extérieur des universités, dans la sphère privée. Vous le savez comme moi, il est facile d'en appeler à la loi, mais le terrain sur lequel nous devons nous placer, avant toute chose,

de corps intermédiaires. L'UNEF est aujourd'hui la deuxième organisation représentative des étudiants en France. Nous devons donc nous préoccuper des valeurs que l'UNEF porte. Nous avons besoin de l'engagement de tous les étudiants pour proposer des solutions. Nous avons besoin de corps intermédiaires pour définir avec eux quelles réponses sont les meilleures, mais nous devons aussi leur rappeler que l'universalisme n'est pas réservé aux livres d'histoire. C'est une valeur moderne, utile, exigeante : une valeur qui fait la grandeur de notre nation.

Soit vous n'avez rien fait, soit votre discours performatif est tout aussi efficace que pour lutter contre le covid ! Comme dirait le ministre de l'intérieur, votre réponse est un peu molle

Parallèlement, cette ambassade a adressé une lettre à notre groupe sénatorial d'échanges et d'études avec Taïwan. L'ambassadeur de Chine Lu Shaye s'est fermement opposé au déplacement de sénateurs français à Taïwan et a menacé ceux qui s'y rendraient. Comme l'an dernier, à la suite d'outrances similaires, le ministre a de nouveau convoqué ce triste diplomate, dont les saillies donnent une bien piteuse image de la Chine, le grand pays avec lequel nous aimerions avoir d'autres relations. Il a eu raison d'agir avec fermeté. La France et le Sénat ne reçoivent pas de consignes du parti communiste chinois. Pour mener le combat idéologique majeur qui nous oppose à la Chine, l'Europe ne peut qu'être unie, nous disiez-vous en octobre dernier. Grâce aux médias, le monde découvre peu à peu avec effroi l'emprise de la dictature du régime de Pékin sur tout le peuple chinois, avec l'aide des nouvelles technologies. Lundi dernier, pour la première fois depuis la répression de Tiananmen, l'Union européenne a imposé des sanctions aux Chinois ayant commis de graves atteintes aux droits de l'homme au Xinjiang contre la minorité musulmane ouïgoure. En réponse, la Chine a sanctionné dix parlementaires européens et des entités de l'Union européenne. hier entre le ministre et ses homologues européens à Bruxelles, M. Le Drian a-t-il envisagé de prendre de nouvelles dispositions vis-à-vis de Pékin ? Pense-t-il que les conditions sont réunies pour ratifier l'accord commercial de l'Union européenne avec la Chine ?

Je rappelle devant vous l'évidence : les parlementaires français décident librement de leurs projets de déplacement et de leurs contacts. Très bien ! Ses propos inacceptables ont valu

Les polémiques publiques, les tentatives d'intimidation, l'insulte et l'invective contre les élus de la République, les institutions académiques, les chercheurs, les médias et, plus largement, la société civile : tout cela n'est pas tolérable dans notre République et n'a absolument pas sa place dans les relations entre la France et la Chine. concerne les mesures annoncées par la Chine en réponse aux sanctions européennes auxquelles vous avez fait référence, notamment à l'encontre de membres du Parlement européen ou des parlements nationaux, comme le député européen Raphaël Glucksmann, de chercheurs et de diplomates, nous les avons fermement et fortement condamnées. J'en profite pour souligner, comme vous l'avez fait, que c'est la première fois depuis trente ans que l'Union européenne adopte des sanctions à l'encontre de la Chine. Cette décision historique est légitime et nécessaire. Il a été solennellement demandé à l'ambassadeur de Chine de rapporter à Pékin que ce n'est pas en attaquant ceux qui ont dénoncé les violations commises ou en s'en prenant à la liberté académique, à la liberté d'expression et aux libertés démocratiques fondamentales que la Chine répondra aux préoccupations légitimes exprimées sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang. S'agissant de nos relations commerciales, la Chine est un partenaire économique incontournable à l'échelle mondiale, mais nos relations ne doivent ni se faire au détriment de nos principes, de nos valeurs et du modèle de société que nous défendons, ni être exemptes de réciprocité.

que les dix ressortissants de l'Union européenne sanctionnés et leurs familles sont dorénavant interdits d'entrée dans la partie continentale de la Chine et dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao.

le Sénat a rejeté la proposition de loi que j'ai déposée avec mon collègue Fabien Gay et le groupe communiste républicain citoyen et écologiste et qui portait sur le statut des travailleurs des plateformes numériques de travail. Cette proposition de loi visait à appliquer le droit social à la relation de travail unissant ces plateformes, telles qu'Uber ou Deliveroo, et leurs travailleurs qui sont dits « indépendants », alors qu'ils sont soumis à leur management algorithmique. L'intégration dans le livre VII du code du travail que nous proposions leur permettait d'accéder à la protection du salariat, tout en renforçant la demande d'une autonomie collective- je parle bien d'autonomie, et non d'indépendance -des travailleurs. En dépit de notre main tendue à votre gouvernement et à tous les groupes de cette assemblée, la droite a voté contre et le groupe socialiste s'est abstenu. Pourtant, les décisions de justice qui se multiplient en Europe nous donnent raison, que ce soit aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, et même en France Toutes confirment notre position : la requalification en salariat fait foi. Je vous le demande donc, monsieur le secrétaire d'État : allez-vous enfin confirmer le statut de salariés de ces travailleurs ?

monsieur le sénateur Savoldelli, les plateformes de mise en relation offrent, il est vrai, des possibilités d'emploi et des services qui sont de plus en plus utilisés et demandés par nos concitoyens depuis quelques années. En cette période de crise sanitaire, nous savons qu'elles permettent aux restaurateurs de développer massivement leur offre de livraison à domicile, ce qui peut compenser pour partie les difficultés auxquelles ils font face. Il est cependant Il est cependant nécessaire que ces nouvelles formes d'emploi ne se développent pas au détriment des conditions de travail et de rémunération des travailleurs indépendants qui y ont recours. Le Gouvernement est convaincu, comme vous, ... Moins que nous ! ... et sans doute comme l'immense majorité des sénateurs, que seul un dialogue structuré entre les plateformes et les représentants légitimes des travailleurs indépendants permettra de rééquilibrer la relation commerciale en faveur de meilleures conditions de travail. La loi d'orientation des mobilités habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les modalités de représentation des travailleurs indépendants des plateformes et les conditions d'exercice de cette représentation. Le Premier ministre a chargé l'ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin, d'une mission visant à préciser ces modalités de représentation. Son rapport a été remis en décembre de l'année dernière. Élisabeth Borne a, par la suite, confié à trois personnalités qualifiées la responsabilité de mener les travaux de rédaction du projet d'ordonnance, en concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des plateformes et des travailleurs indépendants de ces plateformes. Ces travaux ont été menés en tout début d'année, et les préconisations présentées au groupe des partenaires sociaux le 12 mars dernier. Nous avançons ! Le projet d'ordonnance sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'État, en vue d'une adoption par le conseil des ministres au mois d'avril. Son ambition est de rendre effective la représentation, donc de permettre le dialogue social dans la durée avec ces travailleurs de plateforme. Je crois, monsieur le sénateur, que nous pourrions au moins nous retrouver sur cet objectif de représentativité et de discussion équilibrée au sein de ce nouveau type d'entreprise.

Comment expliquer à une esthéticienne qu'elle doit fermer son salon de beauté quand un coiffeur a le droit d'ouvrir ? Les commerçants, comme les Français, sont prêts à faire des efforts. Mais le Gouvernement doit leur parler clairement, sinon quel sens donner à leur sacrifice ? Vos décisions doivent être logiques et, surtout, équitables. Nous vous attendons aussi sur la question des oubliés du fonds de solidarité. Pourquoi les entrepreneurs qui ont repris un fonds de commerce existant sous statut de holding n'ont-ils aucune aide ? Pourquoi les bars-épiceries n'ont-ils pas une indemnisation suffisante ? Vous avez été saisi de plusieurs questions

Le fonds de solidarité, que nous avons mis en place au mois de mars 2020, a d'ores et déjà accompagné 2 millions d'entreprises ; jusqu'à présent, nous avons décaissé 20 milliards d'euros de soutien auprès des entreprises. Nous sommes le pays européen

ne soient pas des critères discriminants pour l'accès au fonds de solidarité, à tel point que 15 % des entreprises aidées n'ont pas de code APE justifiant de leur éligibilité- nous tenons compte de la réalité de leur activité. Nous avons fait en sorte de prendre en charge les entreprises qui ont des coûts fixes particulièrement élevés. Après des discussions

les modifications que nous avons apportées, associées à la réactivité des services de la direction générale des finances publiques, permettent d'accompagner les commerçants et de faire face à la situation. Nous travaillons aussi avec la Banque de France pour faciliter les conditions de remboursement

La décision de la Turquie de quitter la convention d'Istanbul, premier traité international à fixer des normes juridiquement contraignantes pour prévenir les violences sexistes et obliger les gouvernements à se doter d'une législation réprimant la violence domestique, ainsi que le viol conjugal et la mutilation génitale féminine, a été un Cette décision, prise en catimini par simple décret du président Erdogan, est d'autant plus choquante qu'elle intervient quelques jours seulement après le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Nos pensées et notre solidarité vont aux milliers de personnes qui ont eu le courage de manifester dans plusieurs villes turques contre cette décision brutale, ainsi qu'aux femmes turques, de plus en plus victimes de violences. On estime en effet que, en 2020, quelque 300 femmes turques ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre en constante augmentation ces dernières années.

L'Europe ne peut en effet rester silencieuse ou se contenter de simples communiqués face à une décision qui, de fait, encourage les féminicides. féminicides. Aussi, quelles mesures fortes compte prendre notre pays pour mettre fin à la dérive autoritaire de la Turquie ?

comme l'ont indiqué Jean-Yves Le Drian, Elisabeth Moreno et Clément Beaune samedi dernier, avec beaucoup de force, ainsi que les ministres des affaires étrangères de l'Union européennne lors du Conseil des affaires étrangères de lundi dernier, nous déplorons la décision des autorités turques de se retirer de se retirer de la convention du Conseil de l'Europe dite « d'Istanbul », relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, madame la sénatrice, ce retrait affectera particulièrement et en tout premier lieu les femmes turques,

Cette décision est d'autant plus regrettable que la convention d'Istanbul représente l'instrument international le plus abouti en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et, plus largement, contre les violences faites aux femmes. La France rappelle à ce titre qu'elle continuera de promouvoir et d'encourager l'universalisation de la convention d'Istanbul. La lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles demeure au coeur de nos priorités de politique étrangère. En outre, cette décision marque de nouveau une régression en matière de respect des droits de l'homme en Turquie, qui est d'autant plus symbolique que ce pays avait été le premier pays à ratifier la convention en 2011. D'une façon générale, nous restons très vigilants sur la situation des droits de l'homme et du système judiciaire en Turquie. Les autorités turques ne peuvent pas dire vouloir se rapprocher de l'Union européenne

Le 26 février, à Marseille, il a annoncé l'arrivée de « 300 policiers supplémentaires, dont 100 dès 2021 ». Voilà deux exemples annonçant, à grand renfort de communiqués, l'arrivée d'effectifs dans les quartiers. Une chose m'intrigue Darmanin a des policiers en réserve qui ne sont pas sur le terrain ou, pis encore, à qui leur hiérarchie interdit d'aller dans certains quartiers devenus des zones de non-droit ; soit il prend des policiers de certaines circonscriptions pour les déplacer dans d'autres, déshabillant Pierre pour habiller Paul. Le résultat, c'est l'atteinte à notre liberté au travers d'une insécurité qui explose- en hausse de 20 % dans les villes moyennes, en particulier chez les jeunes. La délinquance violente a augmenté de 407 % en cinq ans à Paris.

le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, sillonne la France et répond aux demandes des élus locaux pour garantir la sécurité des Français. C'est aussi le sens de notre stratégie nationale de prévention de la délinquance. Vous évoquez les violences qui concernent les jeunes

soutenir par exemple les interventions faites dans les écoles avec l'éducation nationale. Nous voulons faire de la prévention et de la répression, car l'une ne s'oppose pas à l'autre. Je serai par ailleurs samedi prochain en déplacement

et de toutes. Je terminerai mon propos en saluant les résultats de la police et de la gendarmerie en ce qui concerne le harcèlement de rue. Il faut conclure. Vous avez voté en 2018 une loi pour verbaliser le harcèlement de rue et garantir la sécurité des femmes, notamment les plus jeunes, particulièrement dans les quartiers difficiles. Avec un numéro vert ? J'ai le plaisir de vous annoncer que plusieurs milliers de verbalisations ont été dressées grâce à l'engagement des forces de l'ordre. vous êtes encore dans les effets d'annonce. Je n'ai rien annoncé ! Cela fait tout de même quatre ans que M. Macron et vous-même êtes au pouvoir. La crise sanitaire ne suffira pas à masquer une réalité qui saute aux yeux des Français.

l'immigration, elle n'est pas gérée et nous laissons entrer chez nous la terre entière. Le virus de la délinquance a atteint le taux d'incidence le plus élevé que l'on ait jamais connu, faute de courage.

Vous dites votre fierté du modèle d'élevage bovin « à la française », extensif, familial, herbager, reconnu comme le plus durable au monde, bien loin des canadiens ou brésiliens, qui concentrent des milliers d'animaux élevés aux antibiotiques, mais qui pénètrent toujours plus les marchés européen et français par le cheval de Troie que constituent les traités commerciaux. Monsieur le ministre, votre soutien est précieux, mais vos actes sont déterminants. Aujourd'hui, la situation des éleveurs, notamment des 80 000 éleveurs bovins, continue de se dégrader. Ils s'enfoncent dans la pauvreté et le désespoir, jusqu'à l'acte ultime, comme l'analyse le rapport de nos collègues Françoise Férat et Henri Cabanel, qui vous a été remis, me semble-t-il, ce matin.

vers les zones à faibles rendements, qui n'ont pas ou peu d'autres options et qui sont déjà les mal-lotis des PAC antérieures. C'est la triple peine ! Ce choix n'est ni celui de la filière ni celui de l'Europe. Est-il donc le vôtre, monsieur le ministre ? En avez-vous mesuré les conséquences humaines, économiques et sociales ? Au-delà, quelle est finalement votre vision de l'avenir de l'élevage en France ?

pour utiliser toutes les doses contenues dans les flacons, quel que soit le vaccin, afin de ne jamais être contraint de jeter les doses surnuméraires. Alors même que nous sommes tributaires des approvisionnements en vaccins, de nombreux médecins semblent ne pas pouvoir récupérer les doses surnuméraires. Plusieurs départements sont confrontés à cette situation ; j'ai été alertée, notamment, par les départements du Maine-et-Loire, de la Savoie et de la Haute-Saône. Le recueil de la dernière dose,

AstraZeneca jetées à la suite de la suspension de la vaccination décidée par le Président de la République, on a le sentiment d'assister à un véritable gâchis, au moment où l'épidémie est sur le point de devenir hors de contrôle

ne serait-il pas possible de favoriser des équipements mobiles, au plus près de la population, avec l'appui des élus locaux ? La parole

en flux tendus. Vous le savez, notre campagne vaccinale dépend beaucoup de la livraison de doses de vaccin à notre pays, et celle-ci va s'accentuer à la fin du mois de mars, avec la fourniture de 10 millions de doses de vaccin Pfizer et

vous : pour sortir de cette crise et de cette pandémie, il faut une vaccination massive ; donc, allons-y, vaccinons, vaccinons !

part, de consolider la coopération franco-allemande, dans la lignée du traité d'Aix-la-Chapelle, et, d'autre part, de concrétiser notre vision d'une défense européenne forte et autonome, sur laquelle il existe, en tout cas en France, un consensus. Néanmoins- je le dis sous le contrôle de mes collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées -, nous observons depuis longtemps, lors de nos nombreuses rencontres avec les parlementaires allemands, que notre vision de l'autonomie stratégique européenne ne semble pas partagée outre-Rhin, ni par le Bundestag ni, d'ailleurs, par la ministre allemande

et d'Airbus Defence and Space, pour révéler au grand jour la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons donc, d'un côté, une France pour qui l'avenir est européen, donc franco-allemand, qualificatif que nous étendons au secteur de la défense, et, de l'autre,

jusqu'où sommes-nous prêts à fragiliser notre base industrielle au service d'un projet politique qui semble, malheureusement, de moins en moins partagé par notre partenaire, ce dont nous nous désolons

vous me donnez l'occasion de faire un point d'étape sur le projet du SCAF, le système de combat aérien du futur, qui est très simple : il faut continuer de préparer les démonstrations technologiques avec nos partenaires, travaux très ambitieux, mais indispensables. Ce programme est emblématique de l'ambition qui nous anime : assurer le développement d'une industrie européenne aéronautique et de défense qui soit à la pointe de la technologie et capable de répondre

sur deux ans ; le second, relatif à la première phase de recherche et technologie, autrement dit au lancement du démonstrateur qui volera en 2026, a été signé en février 2021, pour un montant de 150 millions d'euros sur dix-huit concerne la prochaine phase, le ministère des armées échange avec ses partenaires allemand et espagnol, ainsi qu'avec les industriels, afin de définir les travaux qui se dérouleront au cours de la période 2021-2027 et qui visent bien évidemment à mettre en vol, à cet horizon, Chaque pays prévoit de contribuer à parts égales à cette phase, la France restant meneuse du projet. L'objectif reste bien de notifier, dans le courant de 2021, ces travaux l'ensemble des acteurs partagent cette ambition, ainsi que celle d'assurer une entrée en service opérationnel à l'horizon de 2040. Les discussions industrielles dont vous parliez se poursuivent intensivement nous devons nous assurer d'une répartition équilibrée des travaux entre pays, en respectant la logique du meilleur dans son domaine, seule garantie pour nous de réussir à mener ce programme ambitieux dans l'écoute, la qualité et les délais.

Une analyse de l'actualisation stratégique, lancée au cours des derniers mois en association avec le Parlement, nous amène à tirer toutes les conclusions nécessaires pour agir en conséquence, pour ajuster notre effort et pour mieux orienter nos moyens. Au regard de ces conclusions, nous avons constaté que, d'une manière générale, la loi de programmation militaire, ses ambitions et ses priorités conservent plus que jamais toute leur pertinence.

ce type de régime, le Gouvernement propose et le Parlement dispose, c'est-à-dire que l'exécutif exécute les lois et le Parlement contrôle cette exécution. Je ne vois pas au nom de quoi

s'affranchir du respect de la loi. L'article 7 de la LPM est clair : il doit y avoir une révision. Aussi, madame la ministre, je vous le dis comme je le pense, vous appelez souvent le Gouvernement au rassemblement,

La parole est à Mme Françoise Dumont, pour le groupe Les Républicains.

Sur ce nombre, on estime que, dans plus de 30 % des cas, la réponse apportée consiste seulement en une information ou en un conseil médical. Ainsi, en période normale, presque un appel sur trois sature les plateformes, déjà sous forte tension.

cette durée devrait être inférieure à trente secondes, selon les recommandations scientifiques actuelles, pour assurer le bon traitement des situations de détresse immédiate, notamment de l'arrêt cardiaque. Cette question n'est pas nouvelle, et l'enjeu est bien connu au sommet de l'État, puisque, le 6 octobre 2017, M. le Président de la République, Emmanuel Macron, accueillait des professionnels de la protection civile,

Madame la ministre déléguée, comment accepter ce manque d'ambition, ce manque d'action, en particulier dans la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, alors que la population serait prête ?

comme celle que vous avez mentionnée. En effet, il y a différents avantages à tendre vers un numéro unique. Plusieurs États européens ont d'ailleurs déjà fait le choix d'abandonner leurs différents numéros ; je pense à l'Espagne, au Danemark

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Huissiers,

C'est la première fois que nous allons vous entendre en cette qualité dans notre hémicycle. Au nom du Sénat, je vous remercie de votre présence. Je salue la présence de la nouvelle rapporteure générale de la Cour, Mme Carine Camby, à qui je souhaite pleine réussite dans ses fonctions. La présentation de ce rapport annuel devant notre assemblée s'inscrit dans le cadre de la mission d'assistance du Parlement au contrôle du Gouvernement que la Constitution confie à la Cour.

Le contrôle de l'action du Gouvernement est au coeur de la démocratie parlementaire, et l'année de crise sanitaire que nous venons de vivre dans des circonstances exceptionnelles exige de notre part une vigilance rigoureuse et, naturellement, un contrôle attentif et accru des politiques mises en oeuvre. À contexte exceptionnel, pouvoirs exceptionnels, mais aussi contrôle exceptionnel Je le redis, notre démocratie est vivante, et, en cette période où les voies d'urgence restreignent les libertés, nous avons davantage encore un devoir de contrôle. En 2020, nous avons créé un régime juridique spécial d'état d'urgence sanitaire impliquant ces restrictions de liberté. Nos politiques publiques ont subi les effets de la crise et ont dû se réorganiser dans l'urgence pour s'adapter à la situation sanitaire. Nous avons voté des mesures de soutien aux conséquences financières très importantes, tandis que de nombreux secteurs d'activité ont été touchés par la crise. C'est donc sans surprise que

Quelles insuffisances ou erreurs pourrait-on s'épargner à l'avenir ? Vos travaux ont été menés dans des conditions particulièrement contraintes,

soins critiques, l'hébergement et le logement des personnes sans domicile, ou encore certains opérateurs comme la SNCF. Les résultats de certaines de ces enquêtes figurent d'ailleurs déjà dans la première partie de votre rapport. Vous avez également consacré, cette année encore, une part importante de votre activité à répondre aux demandes d'enquêtes formulées par le Parlement en application des articles 47-2 de la Constitution et 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Vous avez ainsi remis pas moins de six enquêtes à notre commission des finances et deux à notre commission des affaires sociales, ce qui est un motif de satisfaction.

En cette période, notre responsabilité d'éclairer les citoyens me paraît essentielle. Je souhaite que le Sénat prenne toute sa part dans cette tâche et joue pleinement son rôle. Cette responsabilité vous incombe également, tandis que vous tirez comme première leçon de cette année de crise, la question de la trop faible anticipation et de l'impréparation des services publics concernés par la situation sanitaire. Votre travail d'enquête, votre analyse et votre regard nous sont précieux et viennent enrichir les

La publication de notre rapport public annuel 2021 intervient, quant à elle, plus d'un an après le déclenchement de cette crise majeure et sans précédent. Bien évidemment, ce choc a eu d'importantes répercussions sur le fonctionnement et les travaux des juridictions financières- la Cour des comptes, mais aussi les chambres régionales et territoriales des comptes, les CRTC -, comme le rappelle l'introduction générale du rapport public. Les raisons en sont multiples ; il s'agit notamment du confinement des contrôlés, de l'allongement des délais de contradiction pour tenir compte des difficultés

n'ont toutefois pas empêché les juridictions financières de remplir leurs missions, avec succès, me semble-t-il, notamment celles qui ont été accomplies au service du Parlement et qui sont essentielles pour nous. Nous avons réalisé, en 2020, pas moins de 16 rapports à la demande de l'Assemblée nationale et du Sénat, et vous avons transmis au total plus de 300 travaux. En particulier, l'année dernière a permis de vous remettre des enquêtes très attendues, que ce soit sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales- je suis venu la présenter devant la commission des affaires sociales -, les politiques de lutte contre la pollution de l'air ou encore la conduite des grands projets numériques de l'État. Je suis donc très heureux que nous ayons pu, malgré le contexte sanitaire,

La crise née de la pandémie de covid-19 a fait émerger, chez les décideurs comme chez nos concitoyens, de nouvelles réalités et de nouvelles préoccupations. Ces réalités, ces préoccupations, les juridictions financières ne pouvaient pas les ignorer. Nous avons donc fait évoluer nos programmes de contrôles, pour prendre en compte cette situation inédite. Au-delà de nos premières analyses relatives à l'impact de cette crise sur les comptes publics, qui ont été publiées dès le mois de juin de juin dernier, j'ai pris la décision de consacrer une grande partie du rapport public annuel 2021 aux effets et à la gestion opérationnelle de la crise du covid-19. Nous avons lancé, dès l'été, de nouvelles enquêtes pour remplir cet objectif. Ce rapport public annuel est donc le fruit de cette année 2020 si particulière. Il présente deux autres originalités, liées, elles aussi, aux circonstances. Tout d'abord, de façon exceptionnelle, il ne comporte pas de chapitre relatif à la situation d'ensemble des finances publiques.

sur ces questions à quelques semaines d'intervalle. Nous publierons le mois prochain l'ensemble de nos analyses sur l'état des finances publiques, avec les données les plus à jour, à l'occasion de ce rapport. Je serai bien sûr heureux de venir les présenter à votre commission des finances si vous en formulez le souhait. seconde originalité, ce RPA 2021 ne contient pas non plus de partie consacrée au suivi des recommandations pour 2020. Réunir les informations correspondantes aurait en effet nécessité d'interroger les services de l'État et des collectivités locales au cours du second trimestre de 2020,

J'en viens maintenant au contenu du rapport public 2021, qui se divise en deux tomes. Le premier aborde les premiers enseignements de la crise, au travers d'une dizaine de chapitres. Le second tome est consacré, de manière plus habituelle, aux politiques publiques et à la gestion publique. Je commencerai par aborder les enseignements et le contenu du premier tome de notre rapport public. Nous avons choisi ici de traiter de sujets importants par leur ampleur opérationnelle ou par les masses financières en jeu, mais aussi d'approfondir d'autres travaux, pour fournir différents éclairages sur la gestion de la crise du covid-19.

consacrés au service public du numérique éducatif pendant la crise sanitaire ou encore à l'hébergement et au logement des personnes sans domicile mettent ainsi en évidence l'absence de plan de continuité dans plusieurs services publics, que ce soit les établissements scolaires ou certaines administrations d'État en charge de l'hébergement d'urgence, ce qui n'a pas permis de couvrir de façon satisfaisante les besoins de protection des plus précaires au début de la crise. De même, l'appropriation du numérique était encore trop limitée pour permettre le basculement rapide dans l'enseignement à distance généralisé. Nous estimons ainsi que 5 % environ des élèves, soit, tout de même, 600 000 enfants, étaient en rupture numérique lors du premier confinement. Un autre secteur trop peu armé pour affronter une crise qui l'a pourtant placé en toute première ligne est celui des services de réanimation et des soins critiques. Ces derniers constituaient, avant la crise, des activités hospitalières très spécifiques et parfois peu connues du grand public- elles le sont,

car le vieillissement de la population soulèvera quoi qu'il arrive la question de l'augmentation des services de réanimation, avec un redimensionnement des effectifs et une réforme des modalités de financement. L'enquête menée par les chambres régionales et territoriales des comptes sur un vaste échantillon d'établissements de santé implantés dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté permet de corroborer, au niveau territorial, les constats de la Cour. Elle souligne, en particulier, que les incertitudes qui entourent le système de collecte et de remontée d'informations, sur lequel se fondent pourtant des décisions stratégiques nationales, constituent un chantier absolument prioritaire.

derniers se sont fortement mobilisés pour faire face aux conséquences de la crise et ont su faire preuve de réactivité, voire d'innovation. Cela vaut bien sûr pour les administrations et services que je viens de citer, mais aussi pour d'autres politiques. Le chapitre consacré à l'aide au retour des Français retenus à l'étranger pendant la pandémie souligne, par exemple, la mobilisation tout à fait exceptionnelle à la fois du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et d'Air France, qui a déployé des efforts considérables, notamment en comparaison d'autres compagnies nationales. Près de 370 000 personnes ont pu ainsi regagner le territoire français, dont 240 000 directement aidées par le ministère, pour un coût total maîtrisé d'environ 8,5 millions d'euros. Le groupe ferroviaire SNCF a également fait preuve d'une très grande réactivité, en mettant rapidement en place une organisation de crise et des mesures sanitaires pour ses personnels et ses clients, mais aussi en anticipant la reprise de l'activité. La circulation des trains de voyageurs a été assurée, tout comme le transport de fret, orienté en priorité vers les besoins essentiels. Notre rapport public aborde également le fonds de solidarité à destination des entreprises, qui constitue l'un des principaux dispositifs de soutien aux entreprises mis en oeuvre par le Gouvernement, avec l'indemnisation de l'activité partielle et les prêts garantis par l'État. l'État. Son succès a été réel et a permis de limiter les effets de la crise, en distribuant rapidement 11,8 milliards d'euros d'aides à 1,8 million d'entreprises. Le fonds s'est transformé après le premier confinement il est passé d'un outil de soutien aux petites entreprises à un outil d'aide plus global et durable pour des structures de plus grande taille. Mais les principes de son fonctionnement, qui repose sur un traitement largement automatisé des demandes, n'ont pas été adaptés en parallèle. Cela accroît le risque d'un cumul d'aides supérieur au préjudice subi et justifie, à nos yeux, le renforcement des contrôles. Ces risques m'amènent à aborder le troisième enseignement de ce premier tome consacré à la gestion de la crise du covid-19 : son coût financier est son coût financier est évidemment très élevé et remet en cause durablement certains modèles de financement. C'est particulièrement vrai pour la SNCF, qui devra faire l'objet d'un suivi attentif, avec un risque de déficit structurel pour le transport à grande vitesse et le fret. Par ailleurs, la crise née de la pandémie a très durement touché les finances d'autres secteurs, comme le montre le chapitre consacré à l'assurance chômage. Cette dernière, qui avait déjà une situation financière dégradée avant la crise, a pleinement joué son rôle de stabilisateur économique et social depuis son déclenchement, en finançant, conjointement avec l'État, le dispositif exceptionnel d'activité partielle. Conséquence logique, l'assurance chômage présente un déficit historique de plus de 17 milliards d'euros en 2020,

Le secteur culturel a également beaucoup souffert depuis le déclenchement de la crise, comme l'illustre notre chapitre consacré à l'institut Lumière de Lyon. Ce remarquable organisme, présidé par le grand cinéaste lyonnais Bertrand Tavernier et créé dans les années 1980 par les héritiers des frères Lumière,

permettent donc d'avoir un premier aperçu de la manière dont la crise du covid-19 a été gérée, même si, encore une fois, nous ne prétendons nullement à l'exhaustivité et si un grand nombre de sujets doivent être revus. L'année 2020 a également vu l'aboutissement d'autres travaux et enquêtes, dans le vaste champ des compétences de la Cour et des CRTC. J'en viens ainsi au second tome du RPA.

et à l'innovation publique. Ce second tome revient tout d'abord sur deux politiques publiques qui ont connu des évolutions importantes et qui seront amenées à jouer un rôle majeur dans les prochaines années. La première est celle qui est menée en faveur de l'inclusion bancaire et de la lutte contre le surendettement ; elle vise à donner à chacune et à chacun la possibilité d'accéder à un compte bancaire, ce qui est aujourd'hui devenu un impératif pour participer à la vie économique et sociale. Ces dispositifs ont beaucoup progressé, mais ils demeurent perfectibles, d'autant qu'ils sont susceptibles d'être très fortement sollicités dans les mois et années à venir du fait des répercussions économiques et sociales de la pandémie, c'est-à-dire- appelons les choses par leur nom -de la montée de la pauvreté qui va accompagner celle-ci. Leur mise en oeuvre devra donc être renforcée, pour mieux accompagner les personnes en difficulté. La procédure de droit au compte, en particulier, gagnerait à être mieux encadrée. seconde politique publique évoquée est l'innovation de défense, qui sera indispensable pour renforcer notre indépendance stratégique, dans un contexte marqué par l'intensification de la compétition mondiale entre pôles de puissance tels que les États-Unis, la Chine ou la Russie.

comme l'aéronautique et le spatial. Nous recommandons, en particulier, de sanctuariser l'effort de recherche en créant un programme budgétaire d'innovation. Le rapport annuel de la Cour s'intéresse aussi de près à l'action publique dans les territoires,

la logique de Philippe Séguin, non pas par l'intégration statutaire, mais par l'intégration fonctionnelle sans cesse renforcée de la Cour et des chambres régionales. Certains de ces travaux abordent les enjeux locaux du changement climatique et de la préservation de l'environnement. C'est le cas du chapitre sur l'optimisation de l'éclairage public dans les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'enquête de la chambre régionale des comptes montre que le bilan des actions entreprises pour diminuer la consommation énergétique est encourageant, mais que la lutte contre la pollution lumineuse, à laquelle nos concitoyens sont très attentifs, demeure en retrait. Ce chantier implique plusieurs paramètres, comme la puissance émise ou la durée de l'éclairage, dans un contexte de forte évolution technologique. La gestion de l'eau doit aussi tenir compte de nouveaux enjeux, notamment en matière de préservation des milieux naturels, comme le montre le chapitre sur la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Les chambres régionales des comptes se sont également intéressées à la situation des quelque 200 communes qui dépendent fortement de l'implantation d'un casino sur leur territoire. Pour ces collectivités, la présence d'un casino assure des recettes nombreuses, la principale étant le prélèvement sur le produit des jeux, qui peut représenter, pour certaines d'entre elles, plus du tiers des recettes de fonctionnement. Nos travaux révèlent que les communes concernées appréhendent souvent la présence d'un casino comme une sorte de rente de situation, dont la crise sanitaire a dévoilé la très grande fragilité. Nous recommandons donc de mieux protéger leurs intérêts à l'avenir, en renforçant leur expertise juridique. Comme chaque année, le rapport public annuel revient aussi, dans ce second tome, sur différents exemples d'actions et de gestions publiques. Il aborde notamment une question que vous connaissez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, à savoir le cas des réseaux consulaires, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, les chambres de métiers et de l'artisanat, les CMA, ou les chambres d'agriculture. Ces chapitres permettent de mesurer les forces et faiblesses relatives de ces de ces organismes. La structuration des réseaux des CCI et des CMA semble plus aboutie, mais le positionnement des chambres d'agriculture est mieux identifié et reconnu. Ces dernières Ces dernières doivent poursuivre leurs mutations internes en encourageant la fusion des chambres départementales, tandis que les réformes sectorielles déjà conduites pour les CCI et les CMA posent, à terme, la question du maintien de leur financement public. Des choix stratégiques devront également être faits pour d'autres organismes. En particulier, le chapitre sur l'ex-agence du numérique montre que l'héritage de cette dernière doit être consolidé, notamment en matière d'inclusion numérique. Cette politique n'a pas encore donné de résultats probants, puisque 17 % de la population- c'est énorme ! -sont concernés par ce que l'on appelle « l'illectronisme » ; il s'agit de personnes sans compétences numériques de base ou qui n'ont absolument pas utilisé internet au cours de l'année écoulée. D'autres dispositifs présentent un bilan bien plus satisfaisant, comme la French Tech, mais doivent être mieux coordonnés et mieux pilotés. De son côté, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, fait montre d'une implication forte, notamment dans la recherche pour lutter contre les pandémies, mais souffre d'une visibilité réduite, en partie liée au caractère dispersé de ses missions et moyens. Le rapprochement organique de l'IRD avec le CNRS apparaît aujourd'hui nécessaire pour renforcer les leviers d'influence et de coopération de la France en matière scientifique et économique. le rapport public annuel aborde deux politiques publiques au coeur des enjeux économiques et sociaux de notre pays. Il s'agit, pour la première, de l'emploi et de la formation professionnelle, au travers de notre insertion sur le pilotage des acteurs associatifs par le ministère du travail. La crise a accentué les tensions sur le financement de ces associations et mis en lumière l'importance de renforcer leur pilotage et l'évaluation de leurs actions. Une autre politique ô combien essentielle abordée dans ce rapport est la santé, avec un chapitre sur la gouvernance des ordres des professions de santé. Nous nous

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, nous avons choisi d'aborder dans ce rapport public annuel des thèmes variés et concrets, sans nous focaliser sur une politique ou un secteur d'administration en particulier. ce rapport ne vise pas à dresser un constat définitif sur la gestion de la crise. Il s'attache simplement, à ce stade, à partager quelques enseignements pour renforcer notre résilience collective face aux prochains chocs- ils viendront

Je suis assez favorable à ce que cette évolution se confirme dans le temps. Cependant, il faut aller plus loin. Notre programmation 2021 sera également très orientée vers la gestion et les conséquences de la crise du covid-19, pour produire un rapport public annuel 2022 qui sera intégralement- je l'annonce déjà -consacré à ce sujet. Vous nous avez d'ailleurs vous-mêmes commandé des travaux cohérents avec ce choix, que ce soit, par exemple, sur la mise en oeuvre et le pilotage du fonds de relance ou sur les mesures de soutien en faveur de la filière aéronautique. Je puis vous assurer que nos équipes sont déjà au travail pour vous rendre en temps et en heure ces rapports qui, j'en suis sûr, seront très suivis, car les questions soulevées par le Sénat sont très importantes. D'ici là, j'aurai remis au Premier ministre l'audit qu'il nous a commandé sur la stratégie d'évolution des finances publiques à la suite du covid-19. Nos travaux sur la crise s'articulent, bien sûr, avec ceux

la très grande diversité de nos missions, notre grande attention portée au niveau local de l'action publique, que je sais cher à vos coeurs de sénateurs. À cet égard, croyez bien que l'intégration fonctionnelle de la Cour des comptes- je le répète encore une fois -est le coeur du projet que je porte. J'aurai plaisir à vous revoir tout au long de l'année 2021, qui sera, je l'espère, toujours aussi riche de nos échanges et de notre coopération. Vous pourrez en tout cas toujours compter sur la cour et son concours. Monsieur le président, en application de l'article L. 143-6 du code des juridictions financières, j'ai l'honneur de vous remettre le rapport public annuel de la Cour des comptes. Il s'agit de

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, le Premier président de la Cour des comptes présente cette après-midi au Sénat le rapport public annuel. Cette présentation est un moment solennel pour notre assemblée, qui illustre et symbolise l'assistance que la Cour des comptes apporte au Parlement, en application de l'article 47-2 de notre Constitution. Cette année, la remise du rapport public a été quelque peu décalée pour permettre à la Cour d'achever l'instruction de ses enquêtes et de livrer ses analyses sur la gestion de la crise. Le Premier ministre lui a également confié une mission relative à la situation des finances publiques et aux priorités de l'action publique pour l'après-crise, ce qui explique l'absence de sa traditionnelle analyse de la situation de nos finances publiques. Alors que le Parlement débat de la soutenabilité de notre dette publique et que la commission Arthuis vient de rendre ses conclusions, nous serons attentifs aux résultats de ces travaux. Je ne reviendrai pas longuement sur le fait que, au-delà de ce rapport public annuel, la Cour des comptes produit de nombreux autres rapports qui nous sont très utiles. La commission des finances vous entend très régulièrement, monsieur le Premier président, comme ce sera encore le cas, le 15 avril prochain, sur l'exécution du budget de l'État.

venus présenter, au cours d'une audition pour suite à donner, l'enquête sur l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU. D'autres auditions seront organisées avant l'été sur le bilan de l'intégration de la gendarmerie au ministère de l'intérieur et sur la couverture mobile en 4G du territoire. De nouvelles enquêtes sont d'ores et déjà programmées pour être remises au début de l'année 2022, dont l'une, très attendue, concernera la mise en oeuvre du plan de relance et sera suivie par le rapporteur général de notre commission, Ces enquêtes complètent utilement les travaux de contrôle et d'évaluation conduits par les rapporteurs spéciaux tout au long de l'année, lesquels donnent lieu à la publication de nombreux rapports d'information- une vingtaine l'an passé -, en dehors même de la période du printemps. Tous ces travaux ont vocation à nourrir et à éclairer nos débats budgétaires. Le premier tome du rapport public annuel a pour ambition de tirer les premiers enseignements de la crise liée à l'épidémie s'agissant de plusieurs politiques publiques. La Cour fait, par exemple, un premier bilan de la politique d'hébergement et de logement des personnes sans domicile pendant la crise sanitaire. Elle souligne la faible préparation de l'État, qui manquait, avant le mois de mars 2020, d'outils opérationnels de gestion de crise, tout en décrivant l'engagement des opérateurs sur le terrain, lequel a permis, dans une situation critique, d'assurer la continuité des missions. L'hébergement d'urgence ne doit toutefois être qu'un point de passage : c'est sur l'accès au logement, en particulier dans les différentes formes de logement social, qu'il nous faut désormais mettre l'accent. Ce premier bilan nous intéresse particulièrement, puisque notre rapporteur spécial Philippe Dallier travaille actuellement sur le sujet. La Cour analyse, en outre, le déploiement des outils numériques qui ont permis d'assurer une continuité des apprentissages dans le contexte de fermeture des établissements scolaires lors du confinement de mars 2020. Comme l'avait fait notre collègue Gérard Longuet dans son dernier rapport budgétaire, rapport souligne que, malgré un succès global et la mise en oeuvre rapide d'outils numériques à grande échelle, la crise sanitaire a soulevé des problématiques d'inégalités d'accès au numérique. Cet enseignement doit désormais guider la stratégie numérique de l'éducation nationale, en intégrant les acquis et l'expérience de la période de confinement.

La crise a révélé les fragilités structurelles dont souffrait déjà la SNCF avant la pandémie, sources de préoccupations quant aux perspectives financières du groupe. Cette question majeure constitue l'un des axes principaux du contrôle que les rapporteurs spéciaux Hervé Maurey et Stéphane Sautarel viennent d'engager et qui a démarré le 9 mars dernier par l'audition du P-DG Jean-Pierre Farandou. Une étude approfondie du déploiement du fonds de solidarité par la direction générale des finances publiques, la DGFiP, est aussi présentée. Pour la Cour, le bilan intermédiaire est globalement positif la DGFiP a su réagir rapidement et efficacement aux problématiques rencontrées par les entreprises lors du premier confinement, même si elle note la complexité croissante du dispositif, qui vise à répondre à un grand nombre de situations et concerne des entreprises de plus en plus importantes. Ces évolutions sont, de fait, porteuses de risques pour nos finances publiques, et ce d'autant plus depuis les annonces visant à prendre en charge une part substantielle des charges fixes des entreprises des secteurs les plus touchés.

au fonds de solidarité à hauteur de 467 millions d'euros en 2020 a témoigné de la mobilisation exceptionnelle des collectivités territoriales face à la crise. La Cour conteste l'autorisation accordée par le Gouvernement d'imputer ces dépenses en section d'investissement. Une telle décision a néanmoins permis de permettre un haut niveau d'engagement des régions aux côtés aux côtés de nos entreprises, sans compromettre leur propre équilibre financier, leur capacité à investir et ainsi, à prendre part à la relance. consacrés à l'assurance chômage rappellent que la baisse des cotisations, la hausse des dépenses d'indemnisation et le financement d'un tiers du dispositif exceptionnel d'activité partielle ont ont provoqué une explosion du déficit du régime, qui s'est ainsi établi à 17,4 milliards d'euros en 2020. La Cour pose donc la question de la responsabilité que doit prendre l'État dans l'effort de redressement de la trajectoire financière de l'assurance chômage, en évoquant notamment la reprise d'une partie de la dette de celle-ci, qui a atteint 54,2 milliards d'euros à la Les comptes de l'Unédic sont, en effet, affectés par des décisions de l'État auxquelles elle est insuffisamment associée. Comme l'ont déjà souligné les rapporteurs spéciaux Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, cette tendance ne date cependant pas de la crise : elle s'était déjà manifestée de la baisse de la subvention de l'État à Pôle emploi, compensée par une contribution croissante de l'Unédic au financement de cet opérateur. Une clarification s'impose sur ce sujet. Le second tome du rapport est consacré à plusieurs politiques publiques et à leur gestion. J'y relèverai deux éléments. D'une part, l'interrogation de la Cour quant au modèle des réseaux consulaires, que vous avez évoqué. Je pense que certains d'entre nous ne partagent pas tout à fait la position de la Cour. Le rapport remet très clairement en cause le financement par une taxe affectée des deux principaux réseaux consulaires, les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, et les chambres de métiers et de l'artisanat, La Cour les considère comme des prestataires de services, qui devraient être financés par le produit de leurs activités commerciales. Or ils assument des missions d'intérêt général et, au cours de la crise, ils ont accompagné, dans un contexte difficile, un très grand nombre d'entreprises. Le dispositif de financement actuel joue également un rôle de péréquation territoriale qu'il ne faut pas négliger. D'autre part, la Cour se penche sur les politiques de lutte contre le désendettement et en faveur de l'inclusion bancaire, de la LOLF et remise à notre commission en juillet 2017, plusieurs auditions que nous avons organisées et la préoccupation que traduit la proposition de loi de notre groupe sur le plafonnement des frais bancaires. La Cour souligne les difficultés rencontrées par la procédure du droit au compte, en recul depuis qu'elle a atteint son plus haut niveau d'application en 2015, du fait de l'insuffisante simplification des procédures et d'une mobilisation hétérogène des réseaux bancaires. Elle constate la grande hétérogénéité des seuils retenus par les établissements bancaires pour apprécier la situation de fragilité financière. Alors que les nouvelles offres de bancarisation ne font pas l'objet d'un plafonnement des frais et accentuent encore l'exclusion numérique, la Cour cite le « maquis » des frais bancaires et leur difficile appréhension par les clients et par les acteurs. Cette situation plaide pour que notre commission continue à travailler sur ce thème. En conclusion, je veux dire ma satisfaction de voir la Cour des comptes jouer tout son rôle en assistant le Parlement dans son contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques et en répondant aux demandes d'enquêtes formulées par les sénateurs, ceux-ci, dans leurs fonctions législatives

le rapport annuel de la Cour des comptes prend, cette année, une forme très particulière, avec une focalisation sur l'analyse des réponses des pouvoirs publics à la crise sanitaire que notre pays traverse encore. vous êtes en quelque sorte allés à l'essentiel, au plus près du vécu et des préoccupations des Français. Pour autant, l'exercice était délicat, puisque plusieurs commissions et organismes s'étaient déjà donné une mission d'analyse du même ordre. Pour ne parler que du Sénat, notre assemblée a mis sur pied une commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire et de sa gestion. Cette commission, présidée par Alain Milon et dont les rapporteurs étaient Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales, Bernard Jomier et Sylvie Vermeillet, a remis son rapport le 8 décembre dernier.

vous avez bien souvent évité l'écueil de la redite. Le Parlement trouvera donc d'intéressantes pistes de réflexion à la lecture de votre rapport annuel. Je centrerai naturellement mon propos sur les chapitres du rapport qui concernent le plus les domaines de compétences de notre commission des affaires sociales : le champ sanitaire, bien entendu, et celui de l'assurance chômage. S'agissant du volet sanitaire, la commission a pris connaissance avec un très grand intérêt des recommandations formulées par la Cour visant à la réorganisation des services de réanimation. Votre rapport souligne, tout comme le faisait d'ailleurs la commission d'enquête du Sénat, que le chiffre des unités de réanimation en France, rituellement brandi comme l'une des preuves de notre retard structurel par rapport à l'Allemagne, ne tient pas compte des unités de surveillance continue.

Vous vous êtes également penché sur les causes réelles des transferts sanitaires de la première vague, sur les raisons de la faible implication, tout au moins dans un premier temps, des établissements de santé privés et sur les effets largement inconnus des déprogrammations massives d'activités hospitalières et libérales. À cet égard, vous soulignez d'ailleurs très bien, à travers les exemples de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Nouvelle-Aquitaine, que, indépendamment du niveau de présence réelle du virus dans ces territoires au cours de la première vague, les établissements ont procédé à des reprogrammations de soins, notamment chirurgicaux, dans des proportions comparables. Dans certains cas, cette réorganisation a même pu permettre d'accueillir des patients covid venant d'autres régions. Les conséquences de ces réorganisations pour les autres territoires pourraient donc être similaires. Vous concluez en recommandant de « mieux tenir compte des besoins lors de la planification sanitaire Le Sénat, chambre des territoires, vous rejoint évidemment sur ce point. Nous avons d'ailleurs récemment tenté de promouvoir les projets territoriaux de santé lors de l'examen de la proposition de loi censée porter la traduction législative des engagements du Ségur Nous ne pouvons qu'espérer, monsieur le Premier président, que les recommandations de la Cour donneront à cette intention le poids qui paraît encore lui manquer ... Pour ce qui concerne votre recommandation d'augmenter les effectifs des médecins réanimateurs et d'infirmières qualifiées, je constate qu'elle rejoint l'appréciation de la commission d'enquête du Sénat. Celle-ci avait aussi constaté que la difficulté venait de l'évaluation locale des besoins en temps réel et du manque d'efficacité des circuits d'information censés renseigner les gestionnaires de crise sur l'évolution territoriale de l'épidémie à l'hôpital. À cet égard, je note que la Cour n'est pas plus parvenue que notre commission d'enquête à évaluer et à localiser les capacités disponibles dans le secteur privé qui n'auraient pas été mobilisées dans la crise. Nous espérons que le temps permettra d'éclaircir ce point et de préciser la gestion de ces lits, en particulier en cas de crise. À l'invitation de la présidente Catherine Deroche, la Cour des comptes aura d'ailleurs l'occasion de poursuivre ses travaux sur l'organisation des services de réanimation et sur leur modèle de financement au-delà de la première vague épidémique de covid-19. La situation actuelle de ces services, lors d'un confinement intervenant un an après la première crise, pourra sans doute apporter de nouveaux enseignements. Pour ma part, je suis convaincu que, au-delà même des services de réanimation, l'organisation d'un système de santé trop centralisé et trop éloigné des territoires constitue une difficulté qu'il nous faudra résoudre afin de gagner en efficacité.

vous rappelez la situation financière dégradée dans laquelle l'Unédic a abordé la crise, ainsi que les changements en matière de gouvernance qui proviennent de l'attribution à l'assurance chômage de ressources fiscales À cette lumière, vous soulignez que les décisions extraordinaires de l'année 2020 ont été prises par l'État, certes dans un contexte d'urgence, mais sans que les partenaires sociaux, théoriquement gestionnaires de l'Unédic, aient leur mot à dire, malgré l'impact financier considérable de ces mesures sur les comptes du régime. Par conséquent, vous recommandez de préciser les rôles respectifs de l'État et des partenaires sociaux dans la détermination des dépenses, des recettes et, bien sûr, de l'amortissement de la dette. de définir, à la sortie de la crise, la nouvelle trajectoire financière qui s'impose, de statuer sur le niveau et les modalités de reprise d'une partie de la dette partie de la dette et de redéfinir le niveau de participation de l'Unédic au financement de Pôle emploi dans un cadre pluriannuel. La commission vous suit largement sur ces préconisations. À nos yeux, il est nécessaire, en particulier, de sortir de l'ambiguïté en matière de gouvernance. C'est pourquoi un rapport d'information de notre commission, qui sera bientôt suivi d'une proposition de loi organique, propose formellement

il est d'une certaine façon rassurant de retrouver cette échéance classique du printemps qu'est la publication du rapport public annuel de la Cour des comptes. Celle-ci permet à la fois de faire le point sur la situation générale des finances publiques au regard des engagements pris en lois de finances et de mettre l'accent sur la gestion de certaines institutions ou administrations. Je regrette simplement la brièveté du délai imparti- moins d'une semaine -entre la publication du rapport annuel et la tenue de ce débat : elle qui ne permet pas d'effectuer une analyse très approfondie de ses quelque mille pages. rapport public annuel rappelle l'impact exceptionnel de la crise sanitaire sur les finances publiques, avec pas moins de quatre budgets rectificatifs l'année dernière.

Vous soulignez également la faible anticipation de la crise sanitaire. Avec le recul, il est vrai que ce manque d'anticipation apparaît comme un grand défaut de la gestion de la crise, sans doute renforcé par un calendrier politique défavorable. il faut tout de suite mettre en regard la forte mobilisation, dès le début, de moyens budgétaires massifs, rendue possible par la suspension des règles du pacte de stabilité. Le Parlement a été au rendez-vous, malgré des conditions de travail compliquées- comme partout ailleurs -, afin de continuer à faire fonctionner la démocratie et les institutions. Ce rapport revient sur la contribution du service public du numérique éducatif à la continuité scolaire pendant la crise sanitaire. En tant qu'ancien enseignant, je tiens moi-même à exprimer ma solidarité et ma reconnaissance envers le monde éducatif, qui a dû faire face, avec les moyens dont il dispose, à un défi inédit. La réouverture des établissements scolaires après le premier confinement doit aussi être considérée comme une chance, alors

La Cour salue, à juste titre, l'efficacité de sa mise en oeuvre. Le montant des aides et les critères d'éligibilité, souples, ont évolué depuis le début de la pandémie. Les mesures de soutien d'urgence ont un coût budgétaire très important. C'est pourquoi notre salut dépend autant de l'efficacité de la campagne vaccinale, qui permettra de rouvrir progressivement les activités. Gageons que la Cour ne manquera pas de s'y intéresser l'an prochain, lorsque nous aurons davantage de recul.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que les transporteurs doivent réaliser des investissements importants pour la rénovation des infrastructures ou encore la transition énergétique. Un autre secteur très fortement touché est celui de l'hôtellerie-restauration. On ne peut que regretter la fermeture de ces lieux de convivialité depuis des mois, en particulier Je terminerai par la situation des réseaux consulaires, notamment des chambres de métiers et de l'artisanat. Leur rôle a été essentiel avant et pendant la crise. Il l'est aujourd'hui pour accompagner les entreprises dans la sortie de crise. L'effort de réorganisation du réseau depuis la loi Pacte a été très important. À la différence des CCI, les chambres de métiers continuent de voir leur activité augmenter. Mon groupe a récemment formulé des propositions visant à soutenir les travailleurs indépendants et les PME. Elles vont, entre autres, dans le sens du renforcement du stage de préparation à l'installation des artisans et du maintien des centres de formalités des entreprises. On ne saurait assez insister sur l'importance des réseaux consulaires dans le maillage économique du territoire. Ce sont des interlocuteurs de proximité et des interlocuteurs naturels pour les entrepreneurs et les artisans. Le maintien d'un financement public nous paraît ainsi essentiel pour garantir l'équité entre toutes les entreprises sur tous les territoires.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, Henry Kissinger aurait affirmé : « Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon agenda est déjà plein ». Année après année, les responsables politiques du pays ont refusé d'anticiper la survenance d'une crise, que celle-ci soit financière, sociale ou sanitaire. C'est ce que je lis dans le rapport de la Cour des comptes

du manque de réflexion de la période d'avant le covid : jamais, par exemple, n'est paru un rapport sur l'activité de réanimation. Pourtant, la saturation des lits de réanimation ne date pas de la crise sanitaire ! Depuis au moins une décennie, elle est bien connue des personnels médicaux.

Indépendamment d'une éventuelle crise sanitaire, nous savions que nous ne pourrions pas faire face à des besoins de soins accrus avec des moyens en baisse. Or, entre 2013 et 2019, la France a été amputée de 21 000 lits d'hospitalisation. Mes

qui constituent pourtant près des deux tiers des malades hospitalisés dans ce secteur. Concrètement, en 2013, il y avait 44 lits de réanimation pour 100 000 habitants de plus de 65 ans ; à la veille de la crise sanitaire, il n'y avait plus que 37. Sans entrer dans les détails du rapport, nous y trouvons bien d'autres choses que nous savions déjà, notamment que 5 % des jeunes souffraient de défaut d'accès aux outils informatiques et que les 600 000 élèves en rupture numérique ne pourraient pas continuer à étudier. Nous savions que les 300 000 personnes sans domicile, dont 40 000 sans-abri, étaient chaque année plus nombreuses dans cette société confrontée à une exclusion chronique : 10 % de plus par an depuis 2012 Nous savions, comme le souligne la Cour, que l'« absence de préparation opérationnelle », alors même que l'épidémie de H1N1 ou la canicule de 2006 auraient dû permettre une réponse moins confuse, a rendu l'État défaillant

de dépistages. On savait donc, mais on n'en a pas tenu compte. Notre groupe adresse donc ses remerciements à la Cour d'avoir rappelé et précisé ces éléments. Vous l'aurez compris, la gestion de la crise sanitaire s'inscrit dans une situation déjà complexe, sur fond de détresse sociale, de rationnement de services publics et de pression financière sur les collectivités locales. L'afflux de cas n'a pas entraîné un recours aux hôpitaux privés pour combler les carences de l'hôpital public, qui était dépassé : 80 % des patients covid en soin critiques étaient hospitalisés dans le public et seulement 10 % dans le privé lucratif. La fédération représentative de l'hospitalisation elle-même déplore que ces établissements n'aient pas été associés pour soutenir le public, l'exécutif préférant les transferts de patients et les déprogrammations massives. En avril dernier, c'est près d'un acte chirurgical majeur sur deux qui n'a pas été assuré. Concernant le logement de ceux qui n'en avaient pas, à l'heure des successions de confinements, les acteurs de la solidarité sont très critiques : « Tant les objectifs fixés que les outils mobilisés se situent dans la lignée de ceux qui préexistaient

Les rapports des chambres régionales sont souvent quelque peu sévères, parfois à juste titre, avec la gestion des collectivités locales.

le Parlement est un lieu de traditions, et le débat organisé à la suite du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes en est une, qui occupe une place importante. C'est pour moi une première. Je comprends que ce débat, en ces temps de crise sanitaire, ne ressemble en rien à ceux des années précédentes. Au-delà du contexte, l'objet même de notre discussion ne respecte pas vraiment les traditions, car la mouture 2021 du rapport annuel ne traite pas de la situation des finances publiques.

Le rapport annuel dont nous discutons aujourd'hui porte essentiellement sur la gestion de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an. Comme cela a déjà été dit, le principal enseignement formulé par la Cour peut se résumer en quelques mots : manque d'anticipation. Le Premier président Pierre Moscovici l'a clairement dit, le principal enseignement du rapport 2021, c'est la faible anticipation de la crise par la plupart des acteurs publics impliqués.

paru le 25 février de l'an passé, nous met sur la piste. La Cour concluait ainsi son avis sur la situation d'ensemble des finances publiques Il importe que [la trajectoire de finances publiques pluriannuelle] prévoie une réduction du déficit structurel ambitieuse, cohérente avec les règles européennes et ne repoussant pas en fin de période de programmation l'essentiel des efforts à accomplir. En complément, un renforcement de l'effectivité du cadre pluriannuel, pouvant passer notamment par une révision des textes organiques, permettrait de crédibiliser dans la durée un tel engagement. » Autant dire que la Cour des comptes, dans sa comptes, dans sa grande sagesse, n'avait rien vu venir de la mise à l'arrêt de notre économie, du creusement abyssal de notre déficit et de l'explosion vertigineuse de notre dette. Personne ne lui en tient rigueur. Nous pouvons nous appesantir sur le manque d'anticipation des acteurs publics, mais gardons-nous d'en tirer des conclusions bien sévères et très politiques sur ce qu'il fallait faire pour anticiper la crise.

Je crois plus pertinent de débattre de l'avenir, et pour cause : l'enjeu est de reconstruire notre pays, brisé par la crise. Le défi, c'est de dessiner au plus vite une voie de sortie crédible, eu égard aux nouvelles contraintes budgétaires. évidemment, le rapport de la Cour des comptes nous livre des éléments de réflexion aussi nombreux que précieux. Je pense notamment, et de façon non exhaustive, à la baisse du nombre de lits de réanimation, passé de 44 pour 100 000 habitants en 2013 à 37 en 2020 à la forte dégradation du réseau ferroviaire national, qui devra bénéficier, dans les prochaines années, des quelque 4 milliards d'euros alloués à la SNCF dans le cadre du plan de relance aux recommandations sur le pilotage de l'innovation de défense, qui illustre les difficultés de la recherche dans notre pays, laquelle débouche trop rarement sur des innovations de marché déployées à grande échelle. De ces trois exemples, je veux tirer quelques leçons, dont je crois qu'elles pourront utilement guider, au cours des prochains mois, notre action parlementaire. Tout d'abord, l'augmentation de la dépense publique n'induit pas nécessairement l'amélioration du service public- c'est une spécialité française. On le voit, par exemple, avec les équipements de nos hôpitaux publics : malgré l'augmentation continue de nos dépenses depuis plusieurs décennies, la situation n'a cessé de se dégrader et les inégalités territoriales n'ont cessé se creuser. Ensuite, nous aurons besoin de grands projets d'infrastructures pour reconstruire notre pays. La transition écologique doit tirer notre développement économique, et non le freiner. Nous devrons massivement investir dans nos équipements de réseau, qu'il s'agisse du numérique, de l'hydrogène, du souverain, du ferroviaire ou encore de l'internet des objets. Enfin, nous devrons mobiliser toutes les ressources, y compris celles de la société civile, pour enclencher cette reconstruction. Si nous ne voulons pas condamner les générations futures à payer cette crise et sa gestion, nous devons inventer de nouveaux moyens de financer la relance en privilégiant les investissements dans les territoires.

vous avez la parole..

S'il est vrai que c'est dans l'adversité que se révèlent les valeureux, notre service public est un joyau. Dans les administrations centrales, dans les collectivités territoriales, ce sont les fonctionnaires, les agents du service public, qui ont permis au pays de tenir debout. Leur boussole, c'est l'intérêt général, pas les profits à courte vue et encore moins les bénéfices de quelques actionnaires rentiers. Toutefois, les baisses de postes et de moyens, opérées à marche forcée depuis tant d'années,

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, à l'image de l'année qui s'est écoulée, le rapport annuel 2021 de la Cour des comptes est singulier. Il se distingue des précédents rapports par la la crise que nous traversons, par sa structure et, surtout, par son contenu. Comme l'ensemble des juridictions, la Cour des comptes a été contrainte d'adapter ses travaux. La crise sanitaire s'éternise, et son lot de conséquences, en particulier sur l'état des finances publiques, continue de s'aggraver. Les conclusions de la Cour doivent donc nous interroger. Tout d'abord, les enseignements de la crise nous incitent à l'humilité. Ils éclairent les dysfonctionnements qui existent depuis de nombreuses années et que nous devons corriger. Il nous faut prendre conscience qu'un certain nombre de dispositifs sont à revisiter. Le rapport de la Cour pointe en effet des situations financières qu'il nous faut transformer, à commencer par notre système de santé. Pendant la première vague, et encore aujourd'hui- hélas ! -, les déprogrammations massives de soins ont été inévitables. Force est de constater que les services de réanimation étaient mal préparés pour affronter une telle crise. lits de réanimation pour adultes a augmenté de 0,17 % ces six dernières années, cette progression se révèle dix fois plus faible que celle des effectifs de personnes âgées. De plus, le mode de financement des soins critiques a participé indirectement à leur recul progressif au regard des besoins. L'ouverture d'un lit en réanimation médicale suscite un déficit moyen de 115 000 euros par an. réformer le modèle de financement et les capacités d'accueil, pour mieux armer les services de réanimation et de soins critiques. La situation de la SNCF doit également nous interroger. Avec une perte nette de 3 milliards d'euros, la Cour ne voit pas « de perspectives financières favorables pour les deux années à venir ». Comme dans d'autres secteurs, la crise a révélé les fragilités structurelles du transport ferroviaire : mauvais état du réseau, fret peu compétitif, endettement chronique ... Le pacte ferroviaire, voté en 2018, a sans doute pallié certaines de ces insuffisances, qu'il était grand temps de corriger. Toutefois, après tant d'années de négligence et d'abandon, tout ne se résout pas d'un seul coup. De la même manière, la crise nous enseigne que nous devons poursuivre nos efforts pour l'accès au numérique dans le milieu scolaire. La lecture du rapport montre aussi que certains choix ont été bénéfiques pour les finances publiques de notre pays. Affirmer sans nuance que rien n'a fonctionné serait totalement faux. Le fonds de solidarité est un succès dont nous pouvons être fiers. Avec l'indemnisation de l'activité partielle et les prêts garantis par l'État, ce fonds de soutien massif et inédit a limité les conséquences économiques de la crise. Le constat de la Cour des comptes à ce sujet est sans appel appel : « Créé en deux semaines, grâce à la très forte mobilisation de toutes les parties prenantes et au recours le plus large possible à des outils déjà existants, simples et efficaces, il a permis de limiter les effets de la crise par la distribution rapide, 31 décembre 2020, de 11,8 milliards d'euros d'aides à 1,8 million d'entreprises et d'entrepreneurs individuels et indépendants. » De façon progressive, le Gouvernement a su transformer et élargir le fonds de solidarité pour éviter la faillite d'entreprises de plus grande taille, en particulier dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du sport, du tourisme, de la culture culture et de l'événementiel. Nous devrons, demain, faire preuve de prudence pour ce qui concerne l'extinction du dispositif. Mais, à ce jour, le fonds de solidarité a montré son efficacité et continue de le faire. Le coût de certaines mesures a été maîtrisé. C'est le cas de l'aide au retour des Français retenus à l'étranger. Au total, le montant des opérations d'aide au retour a été de 8,5 millions d'euros, soit trente-cinq euros par personne aidée. Les 2 635 ressortissants d'autres pays membres de l'Union européenne pris en charge par des avions affrétés par la France ont permis d'obtenir de la Commission européenne une couverture de 75 % du coût net de ces vols. La solidarité européenne montre ici encore ses bienfaits. Mes chers collègues, oui, la situation est grave. Il serait insensé de le nier. Mais ce bilan est à nuancer : si l'on devait ne retenir qu'une chose de ce rapport, ce serait la réactivité inédite de nombreux organismes publics, qui ont su s'adapter avec une remarquable efficacité. La crise économique des prochaines années appelle à considérer avec beaucoup d'attention les recommandations de la Cour des comptes. Que ce soit en matière d'éclairage public ou de fusion des chambres d'agriculture ou de santé, la gestion des finances publiques doit désormais se heurter au choc économique sans précédent de la crise et à la hausse de l'endettement public. Avec une chute d'activité de plus de 30 % en avril 2020, le PIB français s'est effondré de 8,3 % l'année dernière. C'est un repli inédit depuis 1945. Le déficit de l'assurance chômage est supérieur à 17 milliards d'euros, et le niveau de la dette est estimé, à ce stade, à 120 % du PIB. le Premier ministre a confié à la Cour des comptes une mission relative à la situation des finances publiques. Il a également mis en place une commission sur l'avenir des finances publiques. L'audition de Jean Arthuis, ce matin, par la commission des finances a d'ailleurs été très instructive. Le rapport annuel de la Cour des comptes l'est tout autant. Plus que jamais, nous devons réajuster la gestion et l'évaluation de nos finances publiques. Lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, reprendre la trajectoire des finances publiques engagée en 2017 et les réformes créatrices de croissance doit être une priorité pour notre pays. pays. Il est juste et légitime de s'endetter en temps de crise, mais il faut être capable de retrouver l'équilibre dans les périodes les plus favorables. Tous les gouvernements, sans exception, depuis les années 1970, ont laissé notre solde public Ce gouvernement a contribué à le résorber entre 2017 et 2020, avant que n'éclate la crise. C'est cette trajectoire qu'il nous faudra retrouver.

La dégradation vertigineuse de ces dernières traduit l'ampleur du cataclysme économique provoqué par la crise sanitaire. Encouragés par les banques centrales, les États, et la France en particulier, ont pris des mesures exceptionnelles de soutien, auxquelles est venu s'ajouter l'effet de la récession sur l'encaissement des recettes fiscales.

quant à l'emploi et à la gestion des fonds publics, matérialisée par la publication de son rapport annuel, revêt cette année une importance peut-être plus grande encore. Il est d'ailleurs significatif que sa publication ait coïncidé, jeudi dernier, avec la remise au Premier ministre du rapport de la commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par notre ancien collègue Jean Arthuis, dont nous partageons, dans les grandes lignes, les préconisations. « L'argent magique » n'existant pas, il nous faudra rembourser la dette contractée pendant la pandémie. Nos marges de manoeuvre fiscales étant particulièrement étroites, il nous faudra en priorité actionner le levier de la dépense publique, c'est-à-dire celui des économies budgétaires. À cet égard, l'un des aspects de la crise épidémique qui a été souligné par la Cour dans le tome I de son rapport annuel nous interpelle tout particulièrement : la situation de la réanimation et des soins critiques en général. Les magistrats de la Cour des comptes déplorent « l'impréparation du secteur à affronter une crise sanitaire d'une telle ampleur ». La crise de la covid-19 a mis en lumière les carences de l'hôpital public, spécifiquement l'insuffisance et les grandes inégalités territoriales des capacités d'accueil en lits d'hôpital, qui se sont ajoutées à un manque d'effectifs de médecins réanimateurs, alors que les besoins d'hospitalisation croissent avec le vieillissement de la population. Des besoins concrets d'intervention de l'État dans le secteur de la santé sont apparus, alors que nos dépenses de santé représentent 11,3 % du PIB, soit le plus haut niveau de l'Union européenne, dont la moyenne s'établit à 9,8 %. Alors que nous avons manqué de médecins réanimateurs formés, les comparaisons internationales mises en exergue par l'OCDE indiquent que nous avons le plus fort taux- 34 % -de personnels à l'hôpital n'exerçant pas de fonction médicale. La Cour souligne également le faible recours aux capacités du secteur privé au plus fort de la pandémie et appelle à une coordination nationale des soins critiques, incluant structures publiques et privées. Nous pouvons nous demander si la rhétorique du manque de moyens ne nous aveugle pas en partie, au détriment du problème de leur meilleure allocation. Ce problème de la bonne allocation des moyens est d'ailleurs celui que rencontre globalement l'État dans la définition et la hiérarchisation de ses priorités. concerne le volet social, la Cour des comptes s'émeut de la dérive des comptes de l'assurance chômage, tout en reconnaissant que celle-ci a pleinement joué son rôle d'amortisseur économique et social, en finançant, aux côtés de l'État, le dispositif exceptionnel d'activité partielle déployé massivement au bénéfice des entreprises et des salariés. La forte dégradation de la situation financière du régime qui s'est ensuivie, avec un déficit annuel de plus de 17 milliards d'euros en 2020, ne peut qu'interroger sur la trajectoire financière de ce régime, déjà largement déficitaire avant la crise. Le niveau de l'endettement, passé de près de 37 milliards d'euros à plus de 54 milliards fin 2020, pose la question de son amortissement et de la reprise d'une partie de la dette de l'Unédic par l'État. En outre, la question de la gouvernance du régime, marquée, comme le souligne la Cour, par une confusion des rôles entre l'État et les partenaires sociaux, appelle sans doute à une réforme plus profonde que celle qui a été engagée par le Gouvernement à la fin de 2019, si nous voulons redéfinir une trajectoire financière de retour à l'équilibre. Cette problématique, comme celle des retraites d'ailleurs, peut difficilement être éludée à brève échéance. Encore faut-il surmonter la pandémie et définir clairement les bases d'un pacte social renouvelé. La France se singularise moins par le niveau des dépenses de l'État que par celui des dépenses sociales. Sans remettre en cause leur légitimité, on peut tout de même s'interroger, et cela d'autant plus que leur efficacité est régulièrement mise en doute, en particulier dans les enquêtes de la Cour des comptes. Un autre volet du rapport a particulièrement retenu notre attention : celui qui concerne l'indemnisation des entreprises au titre du fonds de solidarité. Ce puissant instrument a été, et continue d'être, indispensable à la survie d'un grand nombre d'entreprises durement touchées par la crise dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, du sport ou encore de la culture. montant de plus de 15 milliards d'euros ont ainsi été distribuées, un dispositif simple et efficace, à quelque 2 millions d'entreprises et d'entrepreneurs individuels et indépendants, et, comme l'indique la Cour des comptes, avec un taux de fraude très faible. Là où la Cour semble regretter l'évolution du fonds au gré de la progression de l'épidémie, passant d'une logique généraliste à une logique plus sectorielle, nous pouvons au contraire y déceler une opportune malléabilité, ainsi qu'une précieuse capacité d'adaptation de l'État à l'évolution de la crise sanitaire et économique. Toutefois, nous ne contestons pas que la puissance de l'intervention publique, en aval,

de la part d'une multiplicité d'acteurs, le cumul des aides versées à certaines entreprises soit supérieur au préjudice subi. Les membres du groupe Union Centriste, vous le savez, sont particulièrement vigilants à la lutte contre la fraude, qui, en matière d'aides économiques, comme en matière de fiscalité et d'aides sociales, doit être implacable. En ce sens, nous souscrivons aux recommandations de la Cour des comptes visant à ce que l'élargissement du fonds s'accompagne d'une instruction plus exigeante des aides et d'un dispositif renforcé de prévention de la fraude et des sanctions. Bien d'autres thèmes abordés par la Cour des comptes dans ce rapport montrent combien le coût élevé de la crise a remis en cause certains de nos modèles de financement, nous obligeant à les repenser. Ces observations et ces recommandations seront utiles aux réflexions et aux contributions que notre commission des finances compte mener, dans les prochaines semaines, pour la reconstruction de la trajectoire de nos finances publiques sur le long terme. La parole

S'il a toujours été utile à nos travaux de contrôle parlementaire, il s'inscrit, cette année, dans un contexte exceptionnel. Dans son introduction consacrée à la situation des finances publiques, la Cour dresse le lourd bilan de l'année passée : chute : chute du PIB et explosion du déficit public et de la dette publique. Si les chiffres présentés reflètent évidemment l'impact de la crise sanitaire, force est de constater qu'ils s'inscrivent dans la suite d'une situation déjà défavorable pour notre pays.

Nos mauvais résultats sur le déficit et la dette au regard de ceux de nos partenaires européens trouvent une explication. À son arrivée, le nouveau Gouvernement a d'abord fait le choix d'une baisse des prélèvements obligatoires dirigée vers les entreprises et les contribuables les plus aisés. Dans un second temps, il a dû, après le mouvement des " gilets jaunes ", en plus de la suppression progressive, mais non financée, de la taxe d'habitation, revenir sur les hausses de fiscalité énergétique et de contribution sociale généralisée, après le grand débat national, il a décidé une réduction de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes ». Depuis lors, face à la crise sanitaire et à ses conséquences désastreuses pour l'économie, le Gouvernement a davantage fragilisé les recettes fiscales, notamment en ce qu'il a choisi de baisser massivement les impôts de production, privilégiant les grandes entreprises et poursuivant sa politique de l'offre, mais sans jamais envisager d'augmenter, même exceptionnellement, les contributions des plus aisés et des activités gagnantes de la crise. En réalité, cette crise révèle que la politique économique et fiscale menée depuis 2017 a été très largement vaine. Ce sont trois années de perdues

Dans son rapport, la Cour des comptes dresse un constat éclairant sur les conséquences de la tarification à l'activité, qui ont fait de la réanimation une activité structurellement déficitaire, donc souvent reléguée au second plan. Elle estime que la création d'un lit de réanimation entraîne un déficit moyen de 115 000 euros, ce qui a entraîné un recul progressif du nombre de ces lits en dépit des besoins si criants aujourd'hui. Il nous faut maintenant tirer les leçons de cette crise et faire en sorte que nous nous préparions à celles à venir.

l'effort sans précédent de mise à l'abri des personnes à la rue- près de 300 000 -, et la capacité de contenir les contaminations, alors que l'hébergement collectif aurait pu les faire exploser. Dès lors, pourquoi arrêter cette politique, qui, malgré un démarrage difficile, Le surcoût annoncé de 326 millions d'euros pour les places supplémentaires est tout à fait absorbable budgétairement, au vu de l'enjeu. Et je n'aurai pas la mauvaise manière de comparer ce montant à celui qui a été

2017. Nous avons là l'occasion de réaliser un grand progrès. La Cour des comptes le souligne : « L'ensemble de ces mesures exceptionnelles a permis d'éviter une surmortalité des personnes à la rue ou sans domicile. Elles ont conduit à une situation sans précédent, où l'essentiel des personnes sans abri, y compris les plus marginalisées, se sont retrouvées hébergées par l'État. » Pourquoi ne pas poursuivre cet effort ? Ce serait un progrès considérable de notre société. Là encore, puisse le Gouvernement écouter les magistrats de la Cour En tant que rapporteur spécial de la mission budgétaire « Action extérieure de l'État », je ne veux pas manquer l'occasion de souligner la grande efficacité du plan déployé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour rapatrier, au printemps

Je l'ai défendu avec mes collègues socialistes au travers d'une proposition de loi qui n'a pas trouvé grâce aux yeux du Gouvernement, malgré les engagements pris devant les Français depuis 2018. Comme nous, la Cour des comptes dresse le constat que « l'opacité qui entoure les frais occasionnés par les incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement, et l'absence d'information des pouvoirs publics à la fois sur leur montant global et sur leur détail par catégorie de clients et de frais, sont un obstacle à une appréhension correcte de difficultés qui concernent chaque année un quart des clients particuliers et plus de deux millions de clients en situation de fragilité financière. En recommandant de poursuivre les travaux d'évaluation et de suivi des frais d'incidents bancaires, la Cour des comptes met bien cette question au coeur de son rapport- c'est une excellente chose ! Il revient au Gouvernement de s'en saisir et d'avancer sur ce sujet, qui a tant d'importance pour nos concitoyens les plus modestes.

de l'assurance chômage et de l'Unédic, la Cour des comptes recommande de statuer sur le niveau et les modalités de reprise de la dette du régime d'assurance chômage. Les décisions prises en la matière permettront à ce dernier de maintenir les indemnisations futures, ou bien conduiront inéluctablement celles-ci à être revues à la baisse. Dans ce contexte si particulier, le rapport de la Cour des comptes nous invite en réalité à réfléchir aux solutions, en sortant des recettes qui sont toujours les mêmes et des blocages idéologiques qui ont présidé à la politique budgétaire et fiscale menée jusqu'à cette crise. Ces réflexes risquent de resurgir dès après, au détriment de nos politiques publiques, des finances de l'État et de la juste répartition de l'effort.

pour nos compatriotes qui les ignorent largement, de rappeler que, en 2020, l'État a dépensé 461 milliards d'euros alors qu'il a constaté 283 milliards d'euros de recettes, portant le déficit Certes, il était nécessaire de soutenir « quoi qu'il en coûte » l'économie, les entreprises, les ménages et les collectivités. Toutefois, en 2019, les comptes publics faisaient déjà apparaître, en dehors de toute circonstance exceptionnelle, un déficit de 93 milliards d'euros, alors que les recettes atteignaient péniblement 301 milliards d'euros ; les dépenses de l'État étaient financées à hauteur de 23 % par la dette. La dégradation est donc bien antérieure à la crise du covid-19. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques, le HCFP, demandait, en septembre dernier, une nouvelle loi de programmation des finances publiques. semble se dessiner aujourd'hui sur la nécessaire stabilisation de l'encours de la dette autour de 120 % du PIB, afin que celle-ci reste soutenable à terme de quelques années, considérant les risques pour l'économie d'un réel effort de désendettement. Cela impliquerait le maintien d'un certain niveau de déficit, sans doute de l'ordre de 3 %, pour les années à venir. Toutefois, cet objectif même est sujet à caution, compte tenu de la hausse prévisible de 11 milliards d'euros de la dépense publique, dès 2021.

mais à arroser les sables d'une bureaucratie galopante qui vient encore de s'illustrer, ces jours derniers, en prétendant faire face à la crise sanitaire avec des attestations et des normes Que reste-t-il des 50 000 postes de fonctionnaires à supprimer durant le quinquennat ? Rien ! Et si l'on regarde l'investissement public net de dépréciation, celui-ci était proche de zéro en 2015 et en 2016, à un misérable 0,4 % du PIB en 2019. Cette réalité serait celle d'une commune très mal gérée ! L'exemple du Grand Paris Express, investissement le plus rentable en termes de recettes publiques, est emblématique : il n'y a aucune participation du budget de l'État à son financement. Cette situation a, et aura, des conséquences multiples. L'incapacité de l'État à soutenir les conseils départementaux, en première ligne pour faire face aux conséquences sociales de la crise économique accompagnant la crise sanitaire, en est l'une des plus préoccupantes, d'autant que les dépenses sociales représentent aujourd'hui près de 60 % des dépenses de fonctionnement des conseils départementaux. Ces dernières années, les départements avaient pourtant amélioré leur situation financière, grâce à de puissants efforts de gestion et à la dynamique de leurs recettes, principalement les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Ils ont ainsi pu augmenter leurs dépenses d'investissement, dont on connaît l'effet de levier sur l'emploi local. Néanmoins, avec la crise sanitaire revient l'effet de

par les mineurs non accompagnés ; augmentation structurelle des dépenses en faveur des personnes âgées d'environ 3 % ; enfin, et surtout, explosion des dépenses de RSA et de lutte contre la pauvreté, au-delà de 10 % pour 2020. Du fait d'un décalage bien connu entre la dégradation de l'emploi et l'inscription au RSA, ce sera pire en 2021 ! Face à ces difficultés prévisibles, l'État, fidèle à sa ligne de conduite avec les départements, s'est montré largement indifférent 200 millions d'euros pour un maigre fonds de stabilisation ; non-reconduction des avances remboursables sur les DMTO en 2021, alors qu'une quarantaine de départements y avaient eu recours en 2020 ; refus de financer l'augmentation au-delà de 5 % du RSA en 2021

sont les départements qui joueront un rôle crucial en sortie de crise. Leurs investissements sont nécessaires au tissu économique local ; ils devront prendre en charge nos compatriotes toujours plus nombreux à bénéficier du RSA, lutter contre la pauvreté, continuer à prendre en charge toujours davantage de personnes en perte d'autonomie et soutenir les enfants dont les familles sont défaillantes. Ils devront aussi, entre autres, maintenir la qualité de l'accueil des collégiens et la sécurité des routes départementales. Dans ce contexte, il est urgent que le Gouvernement s'engage sur une clause de sauvegarde, pour compenser, au moins au-delà d'un seuil à négocier, ce redoutable effet de ciseaux, faute de quoi il ferait courir le risque à notre pays de voir un élément essentiel de sa cohésion sociale en situation de défaillance.

vous êtes mobilisé. Nos travaux se complètent et s'enrichissent parfaitement ; nous partageons les mêmes attentes : plus de transparence et de pédagogie dans la mise en oeuvre et dans les résultats des politiques publiques, plus d'attention portée au coût et à la qualité des services publics, financés par les contributions, et plus de responsabilisation pour les pour les décideurs publics. Cette année, vous avez décidé de consacrer la première partie de votre rapport à différents thèmes liés à la crise du covid-19 ; cela se comprend parfaitement. Vous avez notamment dressé un bilan des deux principales mesures mises en place pour soutenir les entreprises : le fonds de solidarité et l'indemnisation de l'activité partielle. Permettez-moi, à l'occasion de ce débat, de revenir plus particulièrement sur cette mesure d'urgence prise par le Gouvernement pour éviter la faillite d'entreprises, prévenir les licenciements et soutenir le revenu des demandeurs d'emploi. Le Gouvernement a eu un recours massif à l'activité partielle. Comment pouvait-il en être autrement sauver nos entreprises mises à l'arrêt du jour au lendemain ? Toutefois, ce recours massif et les aides exceptionnelles aux demandeurs d'emploi auront mis à mal le système financier de l'assurance chômage, qui était déjà en déséquilibre, avec une dette de 36,8 milliards d'euros à la fin de l'année 2019.

Nous pouvons nous interroger sur le choix de ne pas avoir fait converger les modalités de rémunération entre le public et le privé. En tout état de cause, ce manque de transparence du Gouvernement pose

statuer sur le niveau et les modalités de reprise d'une partie de la dette ? C'est cette transparence et cette pédagogie qu'il faudra bien poursuivre dans la mise en oeuvre et dans les résultats des politiques publiques. Il s'agit d'un principe fondamental, qui contribue à renforcer la confiance entre responsables politiques et citoyens, mais aussi à construire des politiques publiques plus efficientes et plus proches des besoins des usagers. Mais encore faut-il que nous discutions sur la base de véritables chiffres, en temps réel et en toute transparence. La parole

Cet échange avec vous est absolument fondamental à nos yeux ; tel est le sens de notre mission constitutionnelle d'information : je ne la conçois que comme un moment d'échange privilégié avec la représentation nationale.

il est bon que le débat devant les assemblées suive de très près la remise du rapport public annuel au Président de la République. Deuxièmement, je veux formuler une remarque de méthode, qui est aussi une remarque de fond.

Les CCI n'exercent pas uniquement des activités qui relèvent du secteur ou du service public. Elles ont également des activités de nature concurrentielle, d'expertise et de consultation. La gestion déléguée d'infrastructures publiques, qui faisait partie des activités les plus importantes de certaines CCI, est en perte de vitesse, c'est un fait, et les chambres sont de plus en plus en compétition avec les opérateurs privés.

En tant que Premier président de la Cour des comptes, cette fois, je reviendrai dans vos murs dès la semaine prochaine pour l'examen du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire

deux mois une analyse aussi complète de la situation et des perspectives des finances publiques ? J'en suis persuadé. Nous aurons donc un débat riche et étayé sur ces sujets absolument essentiels pour notre pays, dans la terrible période d'incertitudes que nous traversons.

la relation qui nous lie à votre assemblée et les échanges avec le Parlement sont tout à fait cruciaux pour la belle institution que j'ai aujourd'hui l'honneur de présider. Monsieur

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat.- En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions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

la commission des affaires sociales a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 24 voix pour, aucune voix contre -à la reconduction de M. Jean-François Delfraissy à la présidence du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

crise agit en effet comme un révélateur de dysfonctionnements, de rigidités, supportables par le passé, anachroniques aujourd'hui, mais aussi de solutions qui s'imposent à nous et méritent d'être pérennisées. Souvenons-nous, mes chers collègues, au mois de mai 2020, au sortir du premier confinement, le Président de la République, comme le Premier ministre, identifiait un couple maire-préfet de département, capable non seulement d'assurer de concert la scolarisation des enfants de soignants, de fournir des masques, d'organiser une aide concrète pour les citoyens isolés, mais aussi de prendre part à des décisions locales de confinement et de couvre-feu. Ce binôme s'est imposé par temps d'urgence comme un outil plus opérationnel, attestant d'une décentralisation et d'une déconcentration de fait. de fait. Monsieur le ministre, au quotidien, c'est bien au maire et aux conseillers départementaux que les concitoyens s'adressent pour obtenir des réponses concrètes, de même que c'est le préfet que les élus interrogent pour obtenir des réponses et prendre les décisions locales qui s'imposent. élus, le préfet est un interlocuteur naturel, fin connaisseur des territoires, des leviers et des difficultés de proximité. Plus encore, le couple maire-préfet contribue, par ses réponses à nos concitoyens, à faire accepter, bon an mal an, des mesures de restriction sanitaires. Aussi, nous pensons qu'il est désormais temps que cette décentralisation de fait puisse être pleinement légitimée et, de ce fait, améliorée, généralisée ou adaptée à l'ensemble de nos territoires. Notre droit est-il à la hauteur de cette décentralisation ? Chacun ici a en mémoire l'article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. des lois. » Si, comme le Président de la République l'a déclaré, nous sommes en état de guerre sanitaire, alors les intérêts nationaux commandent bien la mobilisation supplémentaire et élargie des préfets de département. Toutefois, les capitaines, si près du front, sont parfois loin des états-majors. C'est vrai ! Si, compte tenu de notre organisation territoriale, le préfet de département a partagé ses compétences avec le préfet de région, il a, en corollaire, trop souvent perdu la connaissance de l'ensemble des décisions de l'administration déconcentrée,

de notre crise sanitaire, à chacun des élus mobilisés aux quatre coins de régions gigantesques et forcément disparates. Le préfet, lui, le peut. Pour cela, nous disposons également d'un outil réglementaire quelque peu oublié, mais qui porte en germe tout un champ de possibilités, en donnant corps à un trio opérationnel : le maire, le préfet et le conseiller départemental. Sans préjudice des dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration permet en effet au préfet de région de « proposer au Premier ministre une modification des règles d'organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s'adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge Plus encore, la conférence nationale de l'administration territoriale de l'État, qui, je dois le rappeler, oeuvre tout à fait séparément des élus de terrain, a pour sa part toute légitimité pour « proposer au Premier ministre tout projet de modification législative ou réglementaire nécessaire à la modernisation et

nous pensons utile de proposer une approche inédite, de procéder dès à présent à des expérimentations préalablement au vote du projet de loi 4D, afin que le préfet du département soit, au moins dans les départements les plus ruraux, l'interlocuteur décisionnaire auprès des maires et des conseils départementaux qu'il puisse, de la même manière, s'appuyer sur le maillage des sous-préfectures. Nul doute que vous trouverez ici des candidats et des partenaires pour y parvenir. Pour cela,

que peu de préfets usaient de ce pouvoir de dérogation, mais que, dans 80 % des cas, les dérogations avaient été très positives. Il y a là aussi sans doute matière à faire vivre une décentralisation de fait sans plus attendre. Les maires comme les conseillers départementaux, avec le concours de leur préfet, pourront, dans la légalité absolue de leurs actes, être ainsi plus efficaces. En temps de crise, l'appareillage technocratique et le cloisonnement des responsabilités ne sont pas de mise.

Mes chers collègues, pour conclure, je redirai ici notre fierté de travailler avec les grands serviteurs de l'État que sont nos préfets. Ils savent comme nous que la proximité est non un simple principe, mais bien une condition de l'efficacité de nos actions communes. La parole

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous ce soir pour débattre, à la demande du groupe du RDSE, du rôle des préfets à l'heure de la relance et de la mise en oeuvre du plan de relance sur l'ensemble du territoire. Annoncé le 3 septembre dernier, ce plan est doté de 100 milliards d'euros. Il nous permet d'accélérer la transition écologique, de soutenir l'activité économique, d'améliorer notre compétitivité et de renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Au 31 décembre 2020, 11 milliards d'euros ont été dépensés, à destination notamment de la SNCF et des collectivités territoriales- par le biais des mesures de soutien à l'investissement, de compensations de recettes ou d'avances remboursables aux autorités de transports

Dès l'origine, nous avons voulu que la relance soit orientée vers les territoires en associant particulièrement les services déconcentrés de l'État, coordonnés par les préfets. Toutes les dispositions du plan de relance ne peuvent être mises en oeuvre à l'échelon territorial, certaines ayant un caractère purement national. dès que nous le pouvons, nous nous appuyons sur cette expertise déconcentrée et sur les collectivités locales. Le maillage territorial pour la déclinaison du plan de relance est ainsi composé, sous la responsabilité et l'autorité de chaque préfet de département, de l'ensemble des sous-préfets sur leur arrondissement, parmi lesquels est désigné un « référent relance » dans chaque département, qui assure un rôle de pilotage. Dans les départements où cela s'est révélé nécessaire, ce réseau a été complété par trente sous-préfets à la relance recrutés à temps plein, à la suite d'un appel à candidatures ayant permis d'examiner 400 candidatures. Leur rôle, sous l'autorité Leur rôle, sous l'autorité du préfet, est d'assurer le bon déploiement de la relance sur le territoire, d'être des interlocuteurs uniques de la relance dans leur département ou leur région pour informer sur le déploiement du plan et lever tous les obstacles qui pourraient se présenter lors de sa mise en oeuvre. Il leur revient également de promouvoir et de valoriser les dispositions du plan, du plan, de coordonner les différents services et les organismes impliqués. Je pense à la Banque des territoires, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ou encore à Bpifrance. Enfin, et peut-être surtout, les préfets ont pour rôle d'associer les collectivités territoriales à la mise en oeuvre du plan de relance. C'est là une condition de sa réussite. je rappelle tout d'abord le soutien massif que l'État apporte aux collectivités locales en cette période de crise économique et sanitaire. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, 16 milliards d'euros seront très concrètement fléchés vers les collectivités, dans le cadre d'enveloppes régionalisées. Au-delà des soutiens à destination des collectivités, nous avons eu à coeur d'associer les élus dès la conception du plan de relance et dans son déploiement. Afin de les accompagner au mieux dans leurs démarches, ma collègue Jacqueline Gourault et moi-même avons mis au point un guide à destination des maires en particulier. Ce guide complet présente les différents dispositifs, les critères éventuels à remplir, ainsi que le calendrier des mesures du plan de relance. Il en précise également les modalités pratiques de mise en oeuvre. C'est aussi le travail commun réalisé par l'État et les collectivités territoriales qui permettra d'atteindre les objectifs Comme l'a rappelé le Premier ministre dans la circulaire relative à la mise en oeuvre territorialisée du plan de relance : « La territorialisation du plan de relance est un gage d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Elle sera l'un des facteurs de sa réussite, en accompagnant les dynamiques territoriales et en rendant possible la consommation rapide des crédits.

Par ailleurs, ces accords régionaux de relance peuvent être déclinés à l'échelon départemental et intercommunal à travers les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Il est important que cette déclinaison puisse avoir lieu pour accompagner les projets de territoires et cibler les projets prêts à démarrer.

C'est, en somme, un contenant unique des objectifs de chacune des politiques publiques du territoire et des financements octroyés. Depuis le 15 janvier dernier, les préfets font part des périmètres de référence qu'ils arrêtent en concertation avec les élus. Le premier contrat de relance et de transition écologique a été signé à Nantes à la fin Un deuxième a été signé avec la métropole de Lyon. Nombre de collectivités- je pense aux départements de la Charente-Maritime, de la Gironde et de l'Ardèche -ont signé des accords régionaux territorialisés de relance. Notre objectif est que tous les territoires soient couverts par un CRTE d'ici au 30 juin 2021. C'est ambitieux, mais il nous faut faire vite afin de relancer notre économie.

l'heure, une seule communauté de communes n'est pas intégrée dans un CRTE, sur décision de ses élus. Cette méthode d'association des élus, nous l'appliquons aussi dans la mise en oeuvre concrète du plan de relance. Nous arrêtons le maximum de mesures à l'échelon local.

que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question et que le Gouvernement répond pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires,

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, lors de leur prise de fonctions aux mois de décembre et janvier derniers, plusieurs sous-préfets à la relance, interrogés notamment par des médias locaux, étaient dans l'incapacité de préciser l'enveloppe dont ils disposaient pour gérer la relance, alors qu'ils ont été nommés pour veiller à la mise en oeuvre du plan. Si les préfets à la relance gèrent les crédits, quelle est alors la place des élus locaux, qui, eux, pourraient garantir une répartition égalitaire dans nos territoires ?

Cela porte à confusion pour les élus et complique évidemment la participation financière de l'État, tout en privilégiant les plus grandes collectivités. De surcroît, la transparence doit être de mise dans le processus de décision. Dans ce cadre, la publicisation des réponses de l'administration est importante, notamment afin de contrôler les deniers publics et d'évaluer les choix de politique publique. Monsieur le ministre, quelles sont les consignes du Gouvernement pour garantir

une collectivité locale ou un échelon déconcentré. MaPrimeRénov'ou les primes à la conversion du parc automobile sont des politiques nationales qui s'appliquent de manière indistincte sur le territoire en fonction de la demande et des projets des ayants droit.

qui peuvent être articulés avec les moyens et les politiques mis en oeuvre par les collectivités locales- région, département, ou bloc communal, avec les intercommunalités -, sans qu'il y ait nécessairement de confusion. Enfin, nous veillons chaque fois que nous le pouvons à associer les collectivités locales

950 millions d'euros sont fléchés sur les collectivités locales. Les préfets recevront dans les prochains jours les notifications, département par département, de ce que représente cette DSIL verte- je la nomme ainsi pour la différencier de la DSIL relance du mois de juillet dernier. Nous estimons que ce sera la meilleure façon d'accompagner les collectivités pour la rénovation énergétique.

qu'à la DSIL rénovation énergétique. Par ailleurs, Jacqueline Gourault et moi-même avons exonéré les préfets de la règle de 20 % pour la collectivité maître d'ouvrage, le temps de la relance et pour les projets exceptionnels portés par des collectivités qui n'auraient pas les moyens d'apporter les 20 % nécessaires.

La mise en oeuvre du plan de relance ne reflète pas véritablement cette volonté. En effet, le choix de placer la majorité des crédits sous la responsabilité des préfets va à l'encontre de la volonté et des souhaits des élus locaux. Il témoigne même d'un manque de confiance envers les territoires, les collectivités se retrouvant souvent contraintes par la préfecture dans l'utilisation des crédits alloués par le plan de relance. De plus, en l'absence de processus clair, précis et transparent, malgré la circulaire envoyée aux préfectures, nous remarquons la diversité des méthodes appliquées par les préfets sur l'ensemble du territoire national. Certains font le choix d'associer et d'informer régulièrement les élus et les parlementaires du territoire, tandis que d'autres limitent ces échanges au minimum. Ainsi, dans mon département, et ce n'est pas un cas isolé, le comité départemental ne s'est réuni qu'une seule fois,

D'autres réunions ne portent que sur des réponses données aux appels à projets, sans débat ni concertation. Dès lors, si la territorialisation paraît nécessaire, les différences de traitement relevées témoignent de l'absence de méthode et de cap. cap. Alors que la mise en place du plan de relance aurait pu être l'occasion d'agir de concert pour construire le monde d'après, notre constat donne lieu à cette question centrale : comment les élus peuvent-ils animer et faire vivre le plan de relance s'ils n'y sont pas réellement associés ?

Régulièrement, Bruno Le Maire et moi-même rappelons à l'ensemble des préfets la nécessité d'associer les élus- parlementaires, maires des communes les plus importantes ou qui structurent le territoire, présidents d'intercommunalité, élus régionaux et départementaux -à la mise en oeuvre du plan de relance. Monsieur le sénateur, je note que vous êtes un élu du département

la part de l'État pour financer des projets qu'il a choisis, dans le cadre d'une discussion entre l'exécutif départemental, la préfecture de département et la préfecture de région. Cela me laisse tout de même imaginer que le débat entre les élus, au moins départementaux, et l'État a été plus fécond que ne le laisse entendre votre question.

Consigne a été donnée à l'ensemble des services de l'État de simplifier au maximum l'instruction des dossiers. Nous le faisons, tout en respectant un cadre législatif et réglementaire. Certains aspects du cadre réglementaire ou législatif ont pu être allégés, d'autres non ;

Ces deux éléments ont d'ores et déjà un impact. Nous avons ouvert un milliard d'euros de DSIL l'été dernier et 950 millions d'euros avec la loi de finances pour 2021. D'ores et déjà,

le rôle du préfet paraît plus que jamais primordial, tout comme est décisive l'importance d'offrir aux élus locaux un interlocuteur de l'État en phase avec la réalité du terrain. La mise en place du plan de relance a pour but de reconstruire le tissu économique, l'attractivité de nos territoires, du préfet, aidé par un chef de projet dans ce domaine, le sous-préfet à la relance. La tâche du préfet est immense, car devront être mobilisés tous les moyens et l'énergie nécessaires pour réinventer la réindustrialisation, l'énergie, la relocalisation, le soutien à l'innovation. ce rôle de développeur en faveur des entreprises, le préfet doit accompagner de façon pérenne les communes et les communautés de communes dans la revitalisation des centres-bourgs, le maintien des services publics et de la santé, le numérique. Cet accompagnement pour l'aménagement des territoires doit constituer la mission prioritaire du préfet. Pendant les premiers mois de la crise sanitaire, les maires étaient au premier rang. Nous avons pu constater l'efficacité du couple maire-préfet pour adapter les règles en fonction des réalités du terrain. Je ne peux que me réjouir du renforcement du lien préfet-maire. À l'heure de la relance, ce circuit décisionnel pragmatique doit non seulement être maintenu, mais aussi perdurer. Il doit devenir un lien naturel de concertation et de différenciation dans les territoires fragiles.

afin de réclamer que 1 % du plan de relance- un milliard d'euros -soit fléché en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou QPPV. Ces revendications ont été entendues. Le Gouvernement a annoncé qu'un milliard d'euros du plan de relance serait bien consacré à ces quartiers ; des annonces ultérieures sont venues compléter cette somme. Cependant, si nous nous félicitons des moyens supplémentaires accordés, une inquiétude demeure au sujet du suivi et de la déclinaison opérationnelle de ces dispositifs dans les territoires. Les élus locaux

Élisabeth Borne, pour la partie emploi, et Nadia Hai, pour la partie politique de la ville, veillent à la mise en oeuvre de ces crédits et à ce que le fléchage que vous appelez de vos voeux soit respecté. Je ne doute pas

Monsieur le ministre, lors de la séance de questions d'actualité au Gouvernement du mercredi 4 novembre dernier, j'ai demandé à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques des précisions sur l'installation des sous-préfets à la relance. Depuis, les trente sous-préfets à la relance, aux profils jeunes et variés, sont entrés en fonction. En tout, il existe 101 « référents relance ». Ces facilitateurs travaillent avec les administrations et les opérateurs de l'État. Bien que mon département de l'Eure n'ait pas reçu de sous-préfet à la relance, la référente étant la secrétaire générale, j'en profite pour saluer le travail important et remarquable du préfet, Jérôme Filippini, ainsi que des sous-préfets. Plusieurs sujets peuvent bénéficier très concrètement de cette territorialisation et reposent entre les mains du préfet.

comme celui qui concerne les jardins partagés, ou encore volontariat territorial en administration (VTA). Aujourd'hui, plusieurs élus de mon département me font part de leur confusion face à la diversité de modalités et au grand nombre d'interlocuteurs : préfet, sous-préfet, référent ou

de chacune des mesures, les contacts pour postuler et être accompagné, les liens utiles, les critères d'éligibilité et le calendrier des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Je souligne d'ailleurs que la publication du calendrier des appels à projets est le fruit d'une suggestion de la mission parlementaire sur la territorialisation du plan de relance, afin de donner de la lisibilité aux élus ainsi qu'aux acteurs du plan de relance.

L'État ayant connu de nouvelles organisations territoriales, il était nécessaire d'adapter le rôle des préfets dans nos collectivités. La modernisation de la gestion des administrations publiques est venue accroître le sentiment que le préfet était un acteur local comme les autres et qu'il peinait souvent à coordonner les actions territoriales des services de l'État. Cela n'est pas forcément vrai partout, en particulier dans les petites collectivités, comme celle que j'ai l'honneur de représenter. Dans mon territoire, contrairement aux propos de mes collègues, le préfet a à la fois un rôle central dans le pilotage de l'action de l'État et un rôle de partenaire. tout, le travers possible d'un tel positionnement est la tentation d'interférer dans la gestion des affaires locales. Au titre du principe de la libre administration des collectivités, il me semble inconcevable qu'un préfet puisse se prononcer publiquement

déclarant qu'il valait mieux s'occuper de la route, et pas forcément goudronner la piste ; on verrait ça plus tard. Il est donc devenu juge de l'opportunité politique

est à M. Yves Détraigne. Au-delà de la communication intensive des services déconcentrés de l'État à laquelle nous assistons depuis quelques semaines, comment les préfets à la relance sont-ils des facilitateurs ? Raccourcir les délais, alléger les contraintes administratives pour permettre les nécessaires investissements stratégiques sur nos territoires : tels sont les enjeux des plans de relance. exemples sur nos territoires tendent à montrer que certaines administrations déconcentrées n'ont pas abandonné

en premier lieu au préfet de mon département, le Gers, qui oeuvre avec détermination depuis le déclenchement de cette crise profonde, dont nous ne voyons pas le bout. Les fonctionnaires d'État ont le mérite de travailler avec professionnalisme dans l'incertitude, confrontés aux ordres et contre-ordres de l'autorité centrale. une telle difficulté, une communication permanente avec les élus a été instaurée. Elle est utile, mais on ne gère bien que ce que l'on mesure. Il faut donc documenter la situation et ses évolutions pour les différentes composantes de la société. Un premier indicateur Cela permet de mesurer les évolutions quasiment au jour le jour et de pointer les déficiences ou les insuffisances que l'on retrouve peu ou prou partout sur le territoire national. La situation sociale doit aussi être observée, en partenariat avec les conseils départementaux. L'économie, de l'artisan au micro-entrepreneur jusqu'à la grosse entreprise, mérite des représentations spécifiques, que les services de l'État, les conseils régionaux, Pôle Emploi et les chambres consulaires sont en mesure de produire. Un tableau de bord, éventuellement normé, nous serait très utile pour constater la situation et ses évolutions, cerner les points sur lesquels l'action doit être portée ou améliorée, en suivre les effets, etc. Le plan d'action France Relance gagnerait aussi à être suivi de la sorte.

Nous l'avons fait pour le plan de relance. Nous le faisons ministère par ministère sur un certain nombre de politiques publiques, même s'il n'y a pas pour l'instant de site récapitulant l'intégralité des travaux de l'État dans tous les départements. Cela n'existait pas avant la crise du covid et c'est toujours le cas

des difficultés rencontrées sur le terrain, disposent d'une expertise comptable utile à la pérennité des entreprises en souffrance.

Par exemple, le fonds de premier secours mis en place par la région et le tribunal de commerce des Hauts-de-France a permis de sauver 3 000 emplois grâce à une aide de 5 millions d'euros.

en activité en sortie de crise épidémique et ce que nous pourrons débrancher. Un certain nombre de dispositions du plan de relance ont vocation à poursuivre l'action et l'effet de dispositifs d'aides. Dans un département comme le vôtre, la baisse des impôts de production représente 411 millions d'euros,

Les appels à projets foisonnent. Ce sont des moules trop souvent façonnés à Paris et les acteurs du territoire- entreprises, administrations ou bailleurs sociaux -se contorsionnent pour s'y couler. Pour ma part, je constate que les sous-préfets sont très mobilisés

Les appels à projets servent toujours ceux qui sont les plus réactifs ou les plus structurés et ceux qui entrent dans le moule préétabli, mais pas toujours les projets les plus adaptés à la spécificité de chaque territoire ou les plus innovants. Sur le volet cohésion, plus particulièrement sur l'accompagnement des jeunes, les mesures sont sont parfois en concurrence ou, au contraire, excluent certains profils. Je pourrais ainsi mentionner les nombreux dispositifs d'accompagnement renforcé et personnalisé pour les jeunes, dont la garantie jeunes, le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea),

manque-t-il pas un peu de cohésion et d'animation locale dans tout cela ? Quel rôle est par exemple réservé aux commissions territoriales emploi-formation, qui sont coprésidées par les régions et les préfets, et auxquelles participent les élus locaux ? Est-il envisagé d'évaluer la pertinence et l'efficacité de ce mode opératoire très encadré les appels à projets ou la multiplicité des dispositifs ? Ces derniers peinent à être lisibles pour ceux qui pourraient en bénéficier, voire pour ceux qui les mettent en oeuvre. La parole est à M. le ministre délégué. Madame

répondrai sur le second, car, très sincèrement, ma collègue ministre du travail serait plus à même que moi d'entrer dans la subtilité d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement vers l'emploi relevant de son ministère.

est mise en oeuvre selon les partenariats département par département, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose de crédits d'aide à l'ingénierie. J'étais à Aurillac voilà quelque temps. Le président du conseil départemental s'est vu notifier

Une trentaine de sous-préfets ont ainsi été nommés auprès des préfectures de département ou de région. Ils sont censés s'assurer que les fonds du plan de relance sont acheminés vers les bons acteurs sur le terrain pour que les appels à projets soient utilisés à bon escient sans favoriser les grands groupes et les plus puissantes collectivités. vous connaissez les critiques dont ces sous-préfets à la relance font l'objet. Je souhaite que vous éclairiez le Sénat sur plusieurs aspects. Tout d'abord, que répondez-vous à la remarque selon laquelle ces postes sont redondants avec d'autres postes déjà chargés du développement économique ? Le risque d'un court-circuitage du travail actuel des préfets et sous-préfets est réel, sans compter que les collectivités territoriales restent méfiantes envers ce qu'elles considèrent comme un jacobinisme déguisé. Par ailleurs, le choix du Gouvernement est celui d'une diversification des profils. Cette initiative est destinée à ne pas réserver le pilotage de la relance au corps préfectoral. Reste que nombre de ces sous-préfets, dont la moyenne d'âge est de 30 ans, ont délibérément été recrutés dans des secteurs trop éloignés des problématiques économiques. arrivent dans des dispositifs existants, il est à craindre que beaucoup de temps ne soit perdu dans l'apprentissage des réseaux économiques et dans la connaissance des entreprises sur le terrain.

Monsieur le ministre, pourriez-vous dresser le bilan du recrutement de ces sous-préfets à la relance et nous éclairer sur la plus-value que vous estimez avoir apportée à nos territoires en créant cette fonction supplémentaire ? La parole est à M. le ministre délégué. Madame

expériences de chacun. D'autre part, c'est conforme à ce que nous mettons en oeuvre en matière de gestion de la fonction publique et des ressources humaines de l'État depuis le début de ce quinquennat, avec une volonté de mobilité la fois interministérielle et inter-versants. J'ai eu l'honneur de défendre la réforme de la fonction publique, permettant justement d'abattre bien des blocages et des obstacles à la mobilité, que ce soit entre les ministères ou entre les trois versants de l'administration.

Le préfet pourrait animer, faciliter, être médiateur, mettre en cohérence les politiques publiques de territoire, c'est-à-dire simplifier ce magasin de farces et attrapes qu'est devenu l'État avec ses appels d'offres et autres aides diverses ! Il y

M. Laurent Burgoa. Monsieur le ministre, voilà peu de temps encore, votre gouvernement souhaitait encourager des relations préfet-maire plus étroites. Pourtant, aujourd'hui, à l'heure où se pose la question de la relance, donc de l'attribution des crédits de soutien à l'investissement, certains maires se trouvent face à un mécanisme qu'ils jugent occulte. Comment ne pas les comprendre ? Ces décisions d'attribution sont entre les mains des seuls préfets. Hier, le Gouvernement et la majorité parlementaire jugeaient discrétionnaires et d'un autre temps les dotations d'action parlementaire, c'est-à-dire les réserves parlementaires. Aujourd'hui, des sommes considérables sont entre les mains de hauts fonctionnaires, qui n'ont de comptes à rendre à personne.

Les relations privilégiées que les grandes villes entretiennent avec les préfectures et, surtout, leur importante ingénierie confèrent à ces dernières un avantage certain par rapport aux plus petites communes de France. Monsieur le ministre, les crédits de soutien ne ruissèlent pas jusqu'aux petites communes ! C'est la raison pour laquelle, afin de pouvoir les défendre, mais aussi d'être gage de transparence, donc de confiance envers le processus d'attribution, je vous demande de bien vouloir vous inspirer

Mme Else Joseph. Monsieur le ministre, ces derniers mois, la crise sanitaire a révélé bien des fragilités, des lenteurs et des inadaptations dans l'organisation de notre État et de notre administration. Pourtant, c'est à ce même État que les Français sont attachés. Dans les mois à venir, je l'espère, la question de la relance de notre économie sera posée. Nous avons raté la crise, ne ratons pas la reprise. Nous pouvons faire de la relance l'antithèse de ce qui a été défectueux, en agissant directement, au plus près du terrain. Pour cette raison, les préfets sont aux côtés des collectivités locales, qui ne manquent pas d'expertise pour développer des projets économiques et industriels, comme c'est le cas dans mon département des Ardennes. Il y a moins d'un an, ma collègue Sophie Primas proposait la mise en place de de simplification administrative pour les nouvelles implantations industrielles, autour des préfets et en lien avec les élus locaux. locaux. Elles sont nécessaires pour encourager la relocalisation de notre économie. Les services de l'État doivent faciliter davantage encore les projets locaux. C'est dans ce cadre que l'on peut imaginer une saine articulation,

? Monsieur le ministre, le préfet n'est pas seulement une image d'Épinal de la déconcentration. Il doit aussi être l'incarnation vivante et adaptée de l'État stratège, avec plus d'autonomie et de prérogatives. À ce titre, n'hésitons pas à renforcer ses compétences en matière d'éducation et de santé, sujets que l'actualité rend prioritaires.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel rôle pour le préfet à l'heure de la relance, à un moment où notre société n'a jamais eu autant besoin d'autorité et de clarté ? Le plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans doit permettre de reconstruire le tissu économique local, de renforcer l'attractivité de nos territoires, d'accompagner la transition écologique et de lutter contre la précarité sociale. Une architecture spécifique de dialogue entre l'État et les acteurs locaux a été prévue dans la mise en oeuvre de la territorialisation du plan de relance. Ainsi, deux comités de pilotage et de suivi aux échelons régional et départemental ont été créés. Le choix a été fait de contractualiser les modalités de déploiement du plan de relance par le biais d'un « accord régional de relance », signé entre l'État et la région en parallèle du contrat Un contrat de relance et de transition écologique pourra éventuellement être signé entre l'État, d'une part, et les départements, les EPCI et les communes, d'autre part, pour des projets particuliers cofinancés par ces collectivités. Enfin, le plan de relance distingue trois types d'enveloppes de crédits « d'actions territorialisées » : certaines seront gérées de manière déconcentrée par les opérateurs régionaux, d'autres seront directement placées sous l'autorité du préfet, d'autres enfin pourront être déconcentrées au fur et à mesure. Plusieurs mois après le lancement des premières actions de relance, le constat est sans appel : il est nécessaire d'appeler à une meilleure coordination des efforts de relance. En effet, il est à craindre que la superposition de multiples niveaux de décision, de diverses couches contractuelles et de différents types d'enveloppes ne soit source de confusion et de retards. De même, la double contractualisation avec les collectivités prendra nécessairement du temps. Les collectivités ne sauraient être réduites au seul rôle d'opérateurs de l'État. Elles attendent au contraire une meilleure reconnaissance de leur rôle, central, dans la vie économique des territoires. Pourtant, en dépit des annonces de territorialisation, les financements restent en grande majorité octroyés sur décision des préfets. Les collectivités sont bien sûr largement appelées à cofinancer ces actions, sans avoir néanmoins de pouvoir de codécision sur leurs orientations. C'est donc une organisation très verticale du plan de relance qui se dessine, dans laquelle les crédits ayant vocation à irriguer les territoires seront distribués par le préfet, sans véritable prise en compte de la vision stratégique propre des collectivités. Le Gouvernement doit donc oeuvrer à offrir les clarifications et simplifications nécessaires, sous peine que la territorialisation du plan de relance ne soit pas effective avant plusieurs mois et repousse encore un économique déjà étalé dans le temps. Pour venir en renfort des territoires, le Gouvernement a décidé de déployer des sous-préfets à la relance. L'intention est louable : il s'agit de faire remonter tous les blocages administratifs rencontrés sur le terrain. l'envoi de nouveaux fonctionnaires ne risque-t-il pas de conduire à un court-circuitage du travail des préfets en place et de brouiller la qualité du dialogue avec les élus locaux ? sans compter les doublons avec les commissaires au redressement productif et, surtout, avec les 450 sous-préfets en poste, dont certains ont déjà en charge des domaines particuliers, par exemple la ville ou l'égalité des chances. Enfin, le préfet se heurte toujours à de nombreuses difficultés dans l'exercice de ses différentes missions, malgré les réformes engagées afin d'améliorer son rôle d'animation. La crise de la covid-19 nous a éclairés sur la difficile coordination des services déconcentrés et l'absence de pilotage du millefeuille administratif, en particulier les agences régionales de santé, mais aussi les services locaux de l'ANRU, dont l'autonomie rend complexe la mise en oeuvre des politiques publiques dans nos territoires.

Nous avons pu constater ces derniers mois l'efficacité des gestions de crise dans les territoires dès lors qu'elles réunissent, autour du préfet, l'ensemble des acteurs locaux selon un modèle de. Le Le décret de 2020 accorde aux préfets un pouvoir de dérogation aux normes réglementaires dans sept domaines pour motif d'intérêt général, et en cas de circonstances locales particulières, afin de réduire les délais de procédure et favoriser l'accès aux aides publiques. Cette mesure de simplification sera particulièrement appréciée dans le cadre du plan de relance et permettra aux préfets, attentifs aux difficultés d'application des règles, de s'engager en faveur d'un dialogue à l'échelon local.

heures - Débat sur le thème : « Quelle perspective de reprise pour une pratique sportive populaire et accessible à tous ? » (demande du